Bonsoir. Mes chers collègues, Madame le ministre. La séance est reprise l'ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 23 et 24 mars 2023. La parole est à madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe. Merci madame la présidente. Monsieur le président de la commission des Affaires européennes. Monsieur le rapporteur général aux finances. Monsieur le vice-président de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Mesdames, et messieurs les sénateurs, je je vous suis reconnaissante d'être là ce soir. Dans l'actualité qui est la nôtre. Et bien sûr c'est. En ligne avec nos traditions. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour. Vous présenter échanger comme de coutume avant chaque conseil européen. Les principaux sujets qui seront traités. comme vous le savez, les chefs d'État et de gouvernement se sont déjà réunis une fois au début du mois de février et dans deux semaines, ils se retrouveront. Pour assurer le suivi de notre réponse au sujet qui continue d'être en haut de l'agenda. La guerre en Ukraine reste bien sur le sujet le plus brûlant. Mais il y aura aussi la réponse que l'Union européenne doit apporter à l'infection, une réduction Act. Ainsi qu'aux réflexions sur la réforme de la gouvernance économique européenne. le Conseil européen continuera d'être marquée par des discussions sur la situation énergétique. Et sur les questions migratoires. Et en cela, il assurera le suivi des du Conseil européen des 8 et 9 février dernier. Enfin il échangera sur la conférence de soutien aux populations syriennes et turques frappés par les tremblements de terre du 6 février dernier. Voilà comme vous le savez sur l'ensemble de ces sujets. La situation évolue tous les jours et les positions que je vais vous exposer sont bien sûr encore susceptible d'évoluer à l'aune des événements que vous connaissez et des concertations conduites entre Européens. l'Ukraine hein comme je vous disais restera bien sûr une des principales priorités de ce conseil. Et le Conseil européen condamne rare à nouveau la guerre d'agression de la Russie en faisant référence au soutien apporté à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour une paix juste et durable, qui a été votée le 23 février. Et au plan de paix en 10 points du président Zelensky. Il insistera sur la poursuite de la mise en oeuvre des sanctions à l'égard de la Russie en renforçant la lutte contre le contournement de ces mesures restrictives. Il appellera à poursuivent les travaux sur la lutte contre l'impunité. En saluant la création du Centre international pour juger du crime d'agression. cette lutte contre l'impunité. Elle doit également concerner les transferts forcés massif. D'enfants ukrainiens. Par la Fédération de Russie. Comme vous l'avez rappelé dans votre proposition de résolution européenne qui a été adopté à l'unanimité par la commission des affaires européennes. Et d'ailleurs cela va cela la figure aussi dans le dixième paquets de sanctions. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Et sur le sujet de l'Ukraine. Il est extrêmement important que nous restions très unis et fermes sur les messages qui sont envoyés par la France. Et en accueillant dans cet hémicycle le 1er février dernier, le président de la Rada ukrainienne. Vous avez témoigné du soutien indéfectible de de la France à l'Ukraine. Le Conseil européen reviendra aussi sur les travaux concernant l'achat la livraison et la production de munitions au niveau européen. Sur ce point très précis, les travaux sont encore en cours et la question sera abordée en détail au Conseil conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la défense le 20 mars prochain. nos sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des 27 de réitérer leur engagement en faveur de la reconstruction de l'Ukraine. Et leur souhait de poursuivre le travail sur le recours aux actifs russes gelés et immobilisé. Enfin le Conseil reviendra sur la poursuite de l'Initiative céréalière de la mer Noire qui nous espérons vivement qu'elle sera prolongée. Voilà une autre partie substantielle du Conseil européen va être va être consacrée aux questions économiques dans toutes leurs dimensions.

Alors d'abord je crois que il faut que nous n'ayons pas peur des mots et que nous assumions que l'Europe. Être un véritable espace puissance et c'est le passage d'un espace économique à un bus, un espace puissance qui, un pic fondamentalement d'ajouter à l'économie, la capacité d'influence. L'influence de l'Union européenne qui découle en partie de son marché intérieur de près de 500 millions de consommateurs et avec son pouvoir normatif, cela lui donne le moyen de peser de façon décisive sur l'organisation des échanges internationaux. Et nous avons fait valoir auprès de la Commission européenne. Notre vision qui est celle d'une politique industrielle extrêmement ambitieuse. Et c'est d'ailleurs ce même objectif que votre commission des Affaires européennes a appelé de ses voeux dans votre proposition de réélu solution du 8 février. Sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2023. Comme nous vous y appelé à une réponse européenne forte à l'adoption de l'inflation, une réduction Act américain. Et à la fois par des outils de défense commerciale et par une nouvelle politique industrielle européenne. cette affirmation de la souveraineté européenne se doit vraiment être notre priorité absolue et elle est la traduction directe du discours de la Sorbonne de 2017. L'inspiration du sommet de Versailles de mars 2022 et de la présidence française du Conseil. Et pour cela nous devons être en capacité de nous fixer des objectifs à horizon 2030 et d'accompagner l'implantation des capacités de production européenne pour répondre à nos besoins stratégiques. Ces besoins stratégiques qui se sont à la fois les matières premières ou les semi-conducteurs. Et évidemment l'idée que ses capacités permettent la réduction des dépendances de l'Union et la réalisation de sa transition écologique. il y a plusieurs leviers, nous en avons un peu débattu lors d'un débat en séance le 8 février dernier. Et je vais les rappeler ici. D'abord simplifier le cadre réglementaire pour l'octroi de permis. Adapter la commande publique et accélérer les procédures d'évaluation de projets par la commission. On pense au piège bien sûr mais aussi à tout ce qui est aide d'État. Flexibiliser les possibilités de financement via les programmes européens afin d'optimiser ses ressources et mobiliser les capacités d'investissements publics et privés. Soutenir une action renforcée pour notre vivier de talents dans ces secteurs clés puisque nous manquons aujourd'hui de main-d'oeuvre dans bon nombre de ces secteurs. enfin en matière commerciale poursuivre un dialogue soutenu avec tous nos partenaires en mobilisant lorsque cela s'avère nécessaire nos instruments de défense commerciale. En complément. Le conseil aura aussi l'occasion d'avoir un échange sur la gouvernance économique de l'Union européenne. Et dans la continuité des échanges en conseil Ecofine hier, il devrait endosser les conclusions relatives à la révision de la gouvernance économique qui ont été adoptés. C'est évidemment une question fondamentale et on nous en avons débattu ici. Il faut que cette. Cette nouvelle gouvernance reflète à la fois la soutenabilité des finances publiques et nous permettent de répondre aux Didier Ferrand défi. Auxquels nous sommes confrontés. Je crois qu'il y a consensus pour dire que le statu quo n'est absolument pas envisageable. Puisque le cadre actuel est inadapté aux défis qui se posent à l'Union. Que l'on parle. À la fois de la transition et de l'indépendance énergétique de la souveraineté industrielle et il est essentiel que pourra à la fois assurer ses investissements et la croissance. Nous soyons d'accord et que le Conseil s'accordent sur des grandes orientations communes. Qui permettent à la fois la différenciation par pays et d'assurer la la crédibilité des trajectoires budgétaires. Et nous souhaitons à ce titre que la Commission puisse rapidement présenter une proposition législative. Sur la situation énergétique. Comme vous le savez, il y aura le conseil aura lieu avant le nouveau conseil des ministres de l'énergie qui aura lieu à Bruxelles fin mars. ce sera l'occasion d'aborder le sujet de la réforme du marché de l'électricité pour laquelle la Commission a présenté sa proposition hier. Et l'objectif est très clair. Il vous l'avez à nouveau rappelé dans votre proposition de résolution du 8 février. Avancée le plus rapidement possible sur ce sujet de façon à pouvoir adapter. Une proposition d'ici la fin de l'année 2023. Évidemment, le but est de pouvoir agir rapidement sur les prix de l'énergie. cette réforme. Qui est évidemment essentiel doit répondre à 2 objectifs d'abord créer un cadre de marché qui apporte une plus grande prévisibilité. Et une visibilité accrue pour les producteurs d'électricité, comme pour les consommateurs. Et garantir des prix plus stable et moins dépendant des cours des énergies fossiles. Ce cas doit également être plus incitatif pour investir dans les énergies décarbonnées. Ce qui va être essentielle pour réduire nos émissions et surtout et aussi pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Le Conseil sera également l'occasion d'aborder les autres enjeux énergétiques en cours de discussion et notamment l'hydrogène ou encore notre état de préparation pour l'hiver 2023 2024. la France sur ce sujet a une position qui n'a pas varié. L'Union doit se préparer le plus en amont possible à l'hiver à venir et notamment concernant notre approvisionnement en gaz naturel. Ce sera un conseil riche, nous allons ensuite passer. Aux questions migratoires. Puisque comme vous savez les 8 et 9 février dernier, le Conseil a rappelé l'importance de renforcer notre action à l'égard des pays tiers, d'origine et de transit. Au moyen de partenariats qu'ils seront mutuellement bénéfique et respectueux des droits de l'homme et des valeurs de l'Union. L'objectif, il est clair, il est de prévenir les départs irréguliers. Il est d'éviter les pertes de vies humaines. Il est de lutter contre les trafics de migrants et de traite des être s'humains. Et puis enfin de favoriser le retour la réadmission et la réintégration durable des personnes qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur notre territoire, notamment celles qui sont non-éligible à la protection internationale. Dans cette optique. Il est essentiel de mobiliser de façon coordonnée. Les instruments à notre disposition. Pour soutenir et aussi responsabilisés nos partenaires en matière de gestion des migrations. Évidemment, nous devons avoir une approche européenne coordonnée pour faire face à la situation actuelle en Méditerranée centrale. Qui est marqué par l'augmentation constante du nombre de personnes tentant de rejoindre l'Union européenne depuis la Libye, la Tunisie et la Turquie. Ce qui conduit à beaucoup trop de drames humains comme nous l'avons tristement vu le 26 février au large des côtes italiennes. En matière de dimension inter-d'immigration. Le Conseil européen a souligné la détermination des chefs d'État et de gouvernement à maintenir le cap des négociations sur le pacte sur l'asile et l'immigration qui est vraiment la boussole entre responsabilité et solidarité. la dynamique qui a été engagé au Conseil et au Parlement dans les négociations doit absolument être préservé pour que nous maintenions il nous arrivions à notre objectif d'une adoption d'ici exactement un an. Enfin, Monsieur le Président Rapin mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez raison d'insister dans une proposition de résolution sur le rôle de l'Agence européenne de frontières et de garde-côtes il les clés et je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en discuter. Et puis il y aura évidemment un point. Et le Conseil reviendra sur les tremblements de terre tragiques qui ont lieu le 6 février et qui ont fait plus de 52.000 morts en Turquie et en Syrie. Le Conseil des 8 et 9 février, avait exprimé ses sincères condoléances pour les victimes, il avait affirmé sa solidarité sans faille avec les populations des 2 pays. Et depuis, l'Union européenne et ses États membres se sont très rapidement mobilisés de façon coordonnée. Pour apporter une aide financière et matérielle et atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. La situation sur place est extrêmement grave les besoins restant à couvrir sont immenses. Il va donc falloir poursuivre et accroître notre solidarité et notre soutien. Et c'est dans cet esprit que la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Organise une conférence des donateurs, le 20 mars à Bruxelles pour mobiliser des fonds de la communauté internationale en faveur des populations sinistrées. Cette conférence permettra d'assurer la bonne coordination de l'aide versée par les différents contributeurs aux différents acteurs, la logistique est difficile comme vous savez. Et il faut que nous arrivions à couvrir de manière efficace les besoins sur le terrain aux côtés des victimes des séismes. Voilà en quelques mots les enjeux de ce Conseil européen. Madame la présidente. Monsieur le président, Mesdames et sénatrices et messieurs les sénateurs, et je ne doute pas que vos questions nous permettront d'éclaircir certains de ces points, si ce n'est tous merci beaucoup. Merci madame la ministre, j'appelle là monsieur Olivier Cadic vice-président de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées à intervenir pour cinq minutes, chers collègues. Madame

Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a à peine plus d'un an, les 10 et 11 mars 2022. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réunissent à Versailles sous présidence française pour un sommet fondateur de notre politique extérieure commune. L'ensemble des États ont pu affirmer à cette occasion leur engagement au service d'une souveraineté européenne, selon la formule défendue par la France depuis plusieurs années. Depuis un an. La guerre se poursuit dans notre voisinage immédiat. Il est dès lors essentiel que l'Union européenne et ses États membres démontrent leur capacité à maintenir leur unité. Il a prouvé leur détermination à court, moyen et long terme. De devenir un acteur géopolitique à part entière dans les relations internationales. À court terme d'abord j'aimerais aborder la dimension européenne de l'aide militaire livrée aux forces ukrainiennes et plus particulièrement la question des munitions. Sur le plan du financement. La mobilisation dès février 2022, de la Facilité européenne pour la paix, pour financer en commun des livraisons d'armements à l'Ukraine est un succès qui a été largement salué. Les cette enveloppe d'aide adoptée à l'unanimité depuis ainsi que son refinancement décidé récemment. Témoignent de l'efficacité et de la pertinence de ce mécanisme. Toutefois, dans l'immédiat l'efficacité de notre soutien militaire commun rencontrent de nouveaux obstacles qui ne sont pas financiers. Je pense en effet aux limites industrielles de notre appareil productif notamment en matière de fabrication de munitions. À la fin du mois dernier le haut représentant Josep Borrell, estimé à 50.000 le nombre de munitions tirées quotidiennement par l'artillerie russe. Quelques jours auparavant, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg avait déclaré publiquement que les forces ukrainiennes utilisent des munitions à un rythme plus élevé que celui de leur production au sein de l'Alliance Atlantique. Madame la secrétaire d'État. Quelles sont, dans ce domaine les leviers dont dispose l'Union européenne pour coordonner la stratégie des États en matière de livraison des munitions à l'Ukraine, voir pour en accélérer la cadence de production. À moyen terme. Ensuite, il est impératif que les preuves que subit actuellement notre continent jouent un rôle de catalyseur pour la constitution d'une base industrielle et technologique de défense européenne autonome. La boussole stratégique européenne adoptée l'année dernière a fait de l'investissement dans la défense, un de ses axes structurants. Mais nous accusons encore un retard difficile à justifier. Seulement 10 18 % de nos dépenses de défense sont aujourd'hui réalisés en commun. Cet émiettement de l'industrie de défense européenne qui nui à notre crédibilité et à notre unité n'est plus acceptable. Il est impératif que nous intervenions avec vigueur pour empêcher que le déclenchement de la guerre en Ukraine n'ait pour conséquence indirecte d'accroître notre dépendance à l'industrie de défense américaine. Quels sont les instruments dont dispose la France pour défendre notre souveraineté industrielle dans le secteur de l'armement. Sur ce sujet. Vous nous donnerez la position de la France sur l'instrument et dire pas de financement d'achat en commun d'armement. Actuellement discuté au Parlement européen. À long terme, enfin il est nécessaire que nous envisagions l'ensemble des conséquences diplomatiques que la guerre en Ukraine aura dans notre voisinage. Plus particulièrement, je pense aux risques de déstabilisation des pays des Balkans occidentaux. L'ouverture des négociations d'adhésion, l'été dernier avec la. L'Albanie et la Macédoine du Nord a témoigné de la volonté de l'Union européenne de faire avancer le processus d'élargissement. Toutefois, il est essentiel que cette volonté se traduisent par des bénéfices concret et surtout immédiat pour les populations concernées. Je tiens à rappeler à cet égard qui s'est écoulé 17 ans entre l'octroi du statut de candidat à l'Albanie et l'ouverture des négociations d'adhésion. Alors que les stat'stratégies d'influence extérieure. Aussi bien russes que turque ou chinoise convergent vers les pays de cette région. Nous devons leur donner des gages de notre engagement en faveur de l'élargissement. À cet égard, il serait utile que vous nous précisiez la position de la France sur la stratégie européenne dans les Balkans. Enfin, alors qu'un second sommet de la communauté politique européenne est annoncé en juin en Moldavie. Pourriez-vous nous dire quel 1er bilan vous vous tirez de cette initiative française au service de l'intégration en Europe des Balkans occidentaux. Je vous en mer. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Après avoir suspendu l'application des règles du pacte de stabilité et de croissance en 2020 pour permettre aux États de mettre mettre en oeuvre les réponses budgétaires qui s'imposer face à la crise sanitaire. La Commission européenne a engagé à partir d'octobre 2021 une réflexion sur la révision de la gouvernance des finances publiques en Europe. Reposant sur les règles d'un déficit inférieur à 3% du PIB d'une dette publique compte tenu en dessous de 60% du PIB. Et de la mise en oeuvre de procédures de coordination entre les États et de correction des écarts la gouvernance prévue par le pacte de stabilité et de croissance et le TSG n'a pas véritablement permis d'assainir les finances de l'ensemble des États membres de l'Union. Plusieurs critiques avaient été adressées aux mécanismes prévus jusqu'ici d'une part il est vrai qu'il s'appliquer de manière uniforme, c'est-à-dire sans véritablement tenir compte des grandes différences de situations qui peuvent exister, tant du point de vue des finances publiques que des capacités des économies. Une approche plus prudente pragmatiques et différenciées peut ainsi apparaître. Souhaitables dans les phases de consolidation. D'autre part, elles étaient sans doute trop complexe puisque reposant pour beaucoup sur des variables économiques difficilement observables et dont l'évaluation fait débat. À l'instar du PIB potentiel et enfin elle n'était pas suffisamment souple pour permettre de différencier les dépenses qui doivent évidemment être maîtrisé de celles qui sont nécessaires pour faire face aux défis d'avenir je veux parler de la transition écologique ou bien encore de la souveraineté en matière par exemple de sécurité ou de formation. Tout en étant particulièrement sensible à ce que les finances publiques des États et plus particulièrement de la France davantage maîtrisé. J'ai salué l'ouverture d'une réflexion de la sur la réforme de la gouvernance budgétaire qui permettraient de l'adapter aux enjeux du XXIe siècle. La Commission européenne a proposé plusieurs pistes d'évolution dans une communication de novembre 2022 qui ont été présentés hier au Conseil des affaires économiques et financières du Conseil de l'Union européenne. Et qui ont été adoptées par ce dernier. Sans revenir sur la règle de limitation des déficits et de l'endettement respectivement à 3% et 60% du PIB. Je l'ai évoqué, la Commission européenne propose notamment de maintenir le cadre commun de surveillance en rendant plus automatique. La mise en oeuvre des sanctions. Elle propose également que les États s'engagent sur des trajectoires pluriannuelle de moyen terme en décrivant leurs cibles budgétaires ainsi que les réformes et investissements envisagés. Elle propose de tenir compte aussi des investissements prévus pour la transition écologique, le numérique et la défense, et enfin de différencier les objectifs prévus pour chacun des États en fonction de la situation de leurs finances publiques. Je note ces propositions qui devraient pouvoir donner lieu prochainement à des initiatives au plan législatif de la part de la Commission européenne l'existence et la bonne application des règles de convergence budgétaire en Europe sont la condition de notre participation à la monnaie unique du et au marché commun. Par ailleurs, je crois que le pragmatisme du Cadre de gouvernance qui est proposé engage la France. Alors que notre endettement s'élève en 2022. Faut-il le rappeler, à près de 3000 milliards d'euros et notre déficit à 4,7% du PIB, le gouvernement doit faire davantage d'efforts. Pour réduire les dépenses publiques à l'horizon 2027. La trajectoire proposée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques n'était à cet égard pas conforme à nos engagements européens. Elle n'aurait d'ailleurs pas davantage été à ce qui découlerait des propositions de la Commission européenne. Il est donc temps d'anticiper et d'agir. Je dirais également un mot de la crise des prix de l'énergie qui depuis son déclenchement a conduit l'État engager des dizaines de milliards d'euros pour contrer les effets à la fois sur les ménages et les entreprises. Ces dépenses sont nécessaires à court terme, même si elles grèvent durablement nos finances publiques et si elles peuvent ne pas toujours paraître à la hauteur, notamment pour soulager nos entreprises les plus fragiles ou les plus exposés. À plus long terme et nous savons tous. Cette situation n'est pas tenable. Pour nous prémunir à l'avenir d'avoir à affronter ce dilemme entre la protection légitime de nos compatriotes et l'emballement incontrôlable de notre dette. Une réforme structurelle du marché électricité est indispensable. Or les espoirs que nous portons sur le projet de proposition qui doit être présenté cette semaine par la Commission européenne devrait malheureusement être déçu. Le gouvernement semble n'avoir pas réussi à faire valoir nos intérêts qui repose sur un mix électrique décarboné et aux coûts de productions faibles cet ajustement des règles du marché de l'électricité ne permettra pas de décorer les les prix du gaz et d'électricité et à la prochaine crise des prix. J'ai bien peur que nous ne soyons à nouveau contraint de prendre des mesures palliatives d'urgence. Fortement coûteuse et certainement moins efficaces. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. J'appelle maintenant monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général monsieur le vice-président, mes chers collègues. Même si l'actualité nationale et est aujourd'hui focalisé sur la réforme des retraites, il nous revient de ne pas perdre de vue l'échelle européenne et les décisions structurantes qui s'annonce à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil européen. Prévue dans huit jours. Une délégation de la commission des Affaires européennes était d'ailleurs hier au siège du Parlement européen à Strasbourg où elle a pu échanger avec près d'une vingtaine d'eurodéputés français de tous les groupes politiques. Vous y étiez aussi, madame la ministre, comme à chaque session du Parlement européen et nous avons été sensibles au fait que vous passiez nous saluer. Nous avons également pu y rencontrer utilement le commissaire, Thierry Breton. Dans la perspective du prochain conseil européen. En effet, l'Ukraine sera assurément au coeur de son ordre du jour. Or, Thierry Breton, nous a confirmé que le conflit était entré dans une phase critique et que les prochaines semaines seraient décisives. Je ne reviens pas sur les propos d'Olivier Cadic, qui vous a suffisamment, à mon avis. Questionné sur. Sur cette question des munitions. je pense que on attend des réponses importantes d'autant que on pourrait imaginer. Que cette situation nous fasse entrer en réelle économie de guerre. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser et vous le préciserai aussi à Olivier Cadic, dans quelle mesure la France pourra contribuer à répondre aux besoins ukrainiens. Au vu de la dépendance en matière de munitions et sur laquelle le Sénat n'a pas manqué d'alerter le gouvernement depuis plusieurs années. Nous sommes par ailleurs très préoccupé sur le sort de la Moldavie. La menace russe d'en faire la prochaine Ukraine est à prendre au sérieux. C'est ce qui vous a conduite à vous rendre la semaine dernière à Chisinau. Où vous avez retrouvé plusieurs de vos homologues pour manifester votre soutien à la présidente Maia Sandu. À l'occasion de la Journée internationale des femmes. Il est effectivement important de donner un site de la substance à la décision du Conseil européen de juin 2022 d'accorder à la Moldavie le statut de candidat à rejoindre l'Union européenne. Chisinau accueillera. En outre, le 1er juin, le 2ème rendez-vous de la communauté politique européenne. La commission que je préside se propose de prolonger au plan parlementaire cette démarche. Et donc. Madame la ministre. Vous pouvez-vous nous apportez votre appui sur un potentiel déplacement que pourrait effectuer. Notre commission dans un cadre vraiment solidaire par rapport au, au Parlement moldave. Le second grand enjeu du prochain conseil européen sera de finaliser la réponse européenne à la une flèche une réduction Act, vous l'avez évoqué, comme convenu en décembre. Le commissaire breton a eu l'occasion de nous en présenter les grands traits hier comme lui nous voyons trop d'entreprises européennes proprement aspiré. Vers les États-Unis. Nous ne pouvons que regretter le retard avec lequel la riposte européenne est arrivé néanmoins sa structuration semble globalement satisfaisante, elle favorisera l'autonomie européenne sur les matières premières critiques, alors que l'Union est aujourd'hui dépendants des importations à 100 pour % pour la moitié, la moitié d'entre elles. Elle prévoit un nouvel assouplissement du régime des aides d'État avec une clause alignement pour prévenir les délocalisations et en complément un futur règlement zéro émission nette destiné à renforcer l'écosystème des technologies propres dans l'Union Madame la Ministre, pouvez-vous nous rassurer sur 2 points. sur la durée de l'assouplissement en matière d'aides d'État prévu pour être temporaire sera-t-elle aussi longue que celle prévue par l'IRA et d'autre part, sur le Champ des technologies zéro émission et technologies nucléaires pourront-elles bénéficier du futur règlement nous souhaiterions aussi savoir si le levier des marchés publics auxquels les États-Unis n'hésite pas à recourir pour soutenir les technologies propres fera partie de l'arsenal européen et si une préférence européenne en la matière sera requis. Enfin, la Commission vient de présenter la dernière brique de la réponse à l'IRA destinée à juguler la hausse des prix de l'énergie, il s'agit de la réforme du marché de l'électricité, le gouvernement s'en félicitent déjà bien qu'elle ne viennent pas sur le principe fondamental de l'Ordre du de mérite. À ce stade, madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que les spécificités des mix nationaux seront bel et bien pris en compte et que les consommateurs en tireront profit sur leur facture énergétique Jean-François Husson. La. De jour en jour nous mesurons en effet dans nos territoires les dégâts de l'inflation pour nos concitoyens. L'Union européenne se doit de les en protéger. Je vous remercie. Madame la. Présidente madame la ministre, mes chers collègues. Plus d'une année s'est écoulée depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ce que l'on redoutait ce produit. Le conflit dure. Il est trop tôt pour parler d'enlisement. Mais on peut certainement déploré un durcissement. Sur le terrain la dureté des combats à Bakhmout illustre en effet une situation très difficile. De plus, doit-on craindre qu'une guerre initialement confinée à l'Europe se mue en un conflit plus générale. Le flou de Pékin sur d'éventuelles livraisons d'armes à Moscou nous interroge. De même que les manoeuvres de Vladimir Poutine pour pousser l'Iran à l'offensive contre l'Occident. Aussi, si j'ose dire. L'Union européenne doit s'apprêter à affûter ses armes. Tout d'abord à ce stade de la guerre, il ne reste plus de place pour l'hésitation. L'Europe doit définitivement s'accorder sur une vision unique si le peuple russe n'est pas l'ennemi, la Russie de Vladimir Poutine l'est devenu. Tant que ce dernier restera au pouvoir, il apparaît difficile de rétablir la confiance. Pour garantir la sécurité collective. Les pays membres de l'Union européenne doivent donc tout se partager les craintes exprimées depuis longtemps par les membres du centre de l'Europe et des pays baltes. À cet égard en tant que présidente du groupe Moldavie du groupe d'amitié France-Moldavie. Je suis inquiète face aux tentatives de déstabilisation de Krishna ou sa présidente Maya Sandu redoute un plan russe visant à troubler son pays qui est, je le rappelle, candidat à l'Union européenne. Dans ces conditions je ne doute pas que le prochain conseil européen réaffirmera comme il l'a fait lors de sa dernière réunion de février dernier son soutien à la fois à l'Ukraine mais aussi à tous ses voisins menacé par l'impérialisme russe. Dans cette perspective, mon groupe soutient la politique de pression collective engagée par l'Europe, notamment le plafonnement des prix des produits pétroliers. Toutes les mesures restrictives adoptées en étroite coordination et coopération avec les partenaires mondiaux, ainsi que les dispositifs anti-contournement qui les accompagnent. Le dernier Conseil européen a exprimé son soutien à la formule de paix en 10 points présenté par le président Zelensky. Au sein du RDSE, nous sommes bien entendu également dans l'attente de la recherche d'une paix négociée, même si je l'ai dit le dialogue avec Moscou est rompu. En attendant, mes chers collègues, nous sommes dans une impasse pour un conflit qui nous savons impacte directement l'économie européenne. Si les prix de l'énergie se tasse un peu la question de l'énergie sera une nouvelle fois à l'ordre du jour du prochain conseil Madame la Ministre comment recevez-vous les propositions avancées hier par Bruxelles sur le marché de l'électricité. On voit bien qu'une vraie réforme de fond promise par la présidente de la Commission s'éloigne de plus en plus, il semblerait que l'on se contente de stabiliser les prix alors qu'il faudrait revoir leur mode de fixation. En attendant, je dois dire que l'on ne peut qu'accueillir favorablement l'idée d'imposer à tous les fournisseurs d'énergie ayant plus de 20.000 clients particuliers des contrats à prix fixe. De même la possibilité pour les États de réduire la facture des consommateurs est également une bonne chose à un moment où nos concitoyens les plus modestes sont pris en tenaille entre les coûts croissants des charges contraintes et les dépenses alimentaires incontournable. Quant aux petites entreprises les protéger contre les fluctuations des des énergies fossiles par un régime de garantie ou un soutien public aux contrats d'achat de combustibles non fossiles constituent aussi une alternative, une initiative de bon sens si toutes ces mesures pour beaucoup conjoncturel mérite d'être soutenue. Il faut que la France renforce sa vision de long terme, c'est une nécessité pour que notre pays retrouve une grande part de souveraineté énergétique. Vous nous avez confirmé Madame la Ministre que le nucléaire faisait bien partie de la réforme proposée par Bruxelles, compte tenu de notre modèle énergétique. Il est évident qu'il paraît difficile de se passer de centrales nucléaires. Pour autant ce maintien de l'atome dans notre mix énergétique ne doit pas empêcher la France de combler le retard qu'il a pris dans le développement des énergies renouvelables. J'espère que la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, tout juste adoptée que mon groupe a soutenu tiendra ses tiendra Pour terminer, je souhaitais souligner la demande du Bureau européen des unions des consommateurs. Qui recommande à l'Union européenne d'interdire les allégations climatique trompeuse sur les aliments tels que ouvrez les guillemets banane climatiquement neutre je Ce bureau a publié une étude, rappelant notamment que la production de tous les aliments et boissons nécessitera toujours l'émission de carbone que ces allégations induisent les consommateurs en erreur attachés aux questions d'étiquetage des aliments. Je souhaite Madame la Ministre que la France soit attentive à cette politique, ainsi qu'à celle de la protection des indications géographiques protégées sur ce dernier point je voulais souligner qu'une approche harmonisée ne doit pas remettre en cause la richesse l'identité et les usages dans nos territoires pour les produits d'excellence comme vous le savez, près de 200 appellation viticole de l'Union européenne se sont inquiétés de la proposition de réforme des règles en matière d'indication géographique. Il serait question d'externaliser des cahiers des charges vers une agence de l'Union européenne, à savoir l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Merci madame la ministre de rassurer nos producteurs et artisans du goût sur ce volet, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent hein. Madame la présidente. Pascale Gruny pour les. Le groupe des Républicains et vous avez 7 minutes, chers collègues.

Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur général monsieur le vice-président, mes chers collègues. Parmi les nombreux sujets qui seront abordés lors du Conseil européen des 23 et 24 mars. Il y aura celui de la compétitivité de l'Union européenne. Cette compétitivité doit être ardue ardemment soutenu que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel. Il en va de l'avenir de nos économies, mais aussi de notre souveraineté. C'est tout l'objet du plan industriel du Pacte Vert qui sera encore au menu des discussions des 27 à Bruxelles et dont l'ambition est claire décarboner notre économie et enrayer notre déclin industriel et il y a urgence. Depuis plusieurs décennies, les pays émergents exerce sur notre industrie une concurrence de plus en plus vives. Y compris dans des secteurs où l'Europe penser qu'elle aurait toujours une longueur d'avance comme l'aéronautique, le nucléaire ou la grande vitesse ferroviaire. À cela s'ajoute une remise en cause permanente de l'organisation collective du commerce international. Pendant que l'Europe s'évertue à respecter à la lettre les règles multilatérales, la Chine continue ses pratiques commerciales déloyales et les États-Unis se réfugie dans un néo-protectionnisme assumé. Le dernier exemple en date, et la loi sur la réduction de l'inflation dite ira qui va concentrer les fonds publics américains sur les produits Made in America, creusant encore un peu plus les écarts de compétitivité et augmentant le risque de délocalisation de nos entreprises vers les États-Unis. Si l'Europe ne réagit pas ce plan américain pourrait selon la Première ministre faire perdre à court terme 10 milliards d'euros d'investissements à la France et entraîné la perte de 10.000 créations potentielles d'emploi. Dans ce contexte, la nécessité de bâtir une politique industrielle au niveau européen n'est plus une option, mais une obligation. Nous devons nous donner les moyens de jouer à armes égales avec nos concurrents en exigeant la réciprocité dans nos relations commerciales en adaptant notre politique de concurrence à la réalité de l'économie du XXIe siècle et en imposant dans nos programmes de subventions des exigences de localisation des approvisionnements et de la production. Certaines clauses contenues dans le projet de règlement pour une industrie zéro émission nette semblerait vouloir aller dans cette direction. Mais tout cela semble encore bien timide, alors qu'il nous faudra affirmer avec force un changement complet de paradigme. De la même façon, comment comprendre au regard du contexte climatique que ce projet de règlement semble vouloir exclure le nucléaire de son Champ d'application. Comment imaginer que demain l'industrie européenne puisse être à la fois compétitive et sobre en carbone, tout en snobant l'atome. L'alliance du nucléaire lancée par Agnès Pannier-Runacher a visiblement encore beaucoup de travail pour que la commission et certains États membres ouvre enfin les yeux sur cette question fondamentale. Le risque de déclassement touche aussi l'industrie agricole. Je voudrais prendre l'exemple de l'industrie sucrière dans l'actualité, révèle la grande fragilité Téréos ça vient d'annoncer l'affaire, fermeture de 2 de ses usines en France. Comment ne pas y voir la conséquence directe de la pression réglementaire croissante sur les moyens de production, de la culture betteravière. Les sur-transpositions nationales et les distorsions de concurrence en Europe aboutissent inexorablement à une baisse continue des surfaces de betterave et fragilise nos outils industriels qui doivent faire face à un environnement toujours plus concurrentiel. Le choix politique d'interdire totalement les néonicotinoïdes à partir de 2018 a conduit toute une filière dans l'impasse. Madame la ministre allez-vous demander l'activation de la réserve de crises agricoles de l'UE pour venir en aide aux producteurs de betteraves affectés par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur les dérogations d'urgence pour les néonicotinoïdes. Je voudrais également évoquer 2 autres sujets sur lesquels je travaille en ce moment avec la commission des affaires européennes du Sénat. D'abord, la création d'un espace européen des données de santé, si l'on souhaite que nos concitoyens autorise l'utilisation de leurs données de santé à des fins de recherche, il faut leur assurer que celles-ci seront protégés et qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres fins. Il est donc indispensable comme l'a demandé. Le Parlement européen que ces données soient hébergés sur le territoire de l'Union ou les États respectent le règlement général sur la protection des données cet hébergement ne suppose également des technologies de pointe que nous devons maîtriser. Pour cela il nous faut absolument investir davantage, de l'dans le domaine du numérique, sans quoi nous condamne rions notre économie à être en permanence dépendants des technologies venus d'ailleurs. La compétitivité des entreprises passe aussi par un système réglementaire favorable à l'investissement. Nous devons donc être attentif à certaines propositions de règlement comme celle qui propose de réviser le système de redevances perçues par l'Agence européenne des médicaments. Il s'agit de s'assurer que certains produits continueront d'être fabriqués et commercialisés sur le territoire de l'Union. Ainsi, la Commission européenne doit présenter à la fin du mois de mars une réforme de la législation pharmaceutique. Nous comptons sur vous pour veiller à ce que celles-ci permettent le développement effectif d'une industrie pharmaceutique innovante sur le territoire de l'Union mais également le maintien d'une industrie produisant des médicaments plus mature afin d'éviter les pénuries que nous connaissons aujourd'hui. Le 2ème sujet concerne la directive sur les travailleurs de plateforme pour laquelle les négociations au Conseil se poursuivent mais semblent patiner. Au vu des divergences. Encore existantes entre les États, plusieurs questions se posent. Est-il légitime d'espérer un accord au Conseil sous présidence suédoise hein comme celle-ci, l'annonce ou plutôt compter sur la présidence espagnole dont la législation nationale et d'avancer sur ce sujet pour faire aboutir ce texte. La France est-elle prête à faire des concessions pour parvenir à un accord. Pour conclure, chers collègues, sur toutes ces questions ayant trait à la compétitivité de l'Union européenne, nous n'avons d'autre choix que de faire preuve de volontarisme. À défaut, l'Europe risque d'être balayée par des concurrents internationaux toujours plus déterminé et conquérant. Nous sommes donc aujourd'hui à la croisée des chemins où nous nous donnons les moyens de continuer à peser dans les affaires du monde où nous devenons un continent sous influence. Je forme le voeu que l'Europe choisissent la voie du sursaut et non celle du Renaud du renoncement. Merci de votre attention. Merci madame la présidente. La parole est à présent à Madame, Colette Mélot du groupe les indépendants et vous avez six minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre. Messieurs les présidents, mes chers collègues. Plus d'un an que les atrocités sont en cours en Ukraine. Plus d'un an que des enfants ukrainiens sont déplacés massivement vers la Fédération de Russie. Ces enfants sont naturalisés, leurs noms sont changés même leur filiation sont modifiés. Ces crimes sont punies par le droit international et je salue le travail fourni par de nombreuses personnes et organisations afin de faire toute la lumière sur ces faits innommables. La commission des Affaires européennes ici au Sénat. À travailler sur une proposition de résolution européenne à l'initiative de mon collègue André Gattolin. Sur une proposition donc. Qui dénonçaient ces transferts forcés. Plusieurs points concerne l'action de l'Union européenne et vont au-delà des actions qui doivent bien sûr continuer à exercer une pression significative sur la Russie. Nous devons collectivement continue à condamner ces faits, il faut l'aider les documenter le plus précisément possible afin que justice puisse se faire en temps et en heure. Le groupe les indépendants et très investi sur la situation en Ukraine. Nous avons fait adopter au Sénat le 7 février dernier à une très large majorité une proposition de résolution exprimant le soutien du Sénat l'Ukraine. Condamnant la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie et appelant auras renforcement de l'aide fournie à l'Ukraine à l'initiative du président Maluret nous y'dénoncions déjà l'enlèvement des enfants et des déplacements forcés la PP reprolonge prolonge ce travail et j'espère Madame la Ministre que la France portera la vision de ces de PPR au Conseil européen. Ce conflit a aussi de fortes répercussions sur les Européens en matière inerte énergétique. Les annonces de la Commission sur son projet de réforme du marché de l'électricité. Marc d'un 1er point d'évolution, c'est le futur des et des Européens qui se dessine. C'est une nouvelle crise majeure qui nous oblige à avancer. Madame la Ministre quels sont les points principaux que vous défendrez au delà du découplage des prix du gaz et de l'électricité qui n'a pas été retenu. Bien qu'il me semble cependant essentiel de plus comment vont se passer des hivers prochain particulièrement concernant les stocks de gaz, sujet dont on doit se soucie dès l'été les citoyens européens ont besoin de prévisibilité face au prix de l'énergie. Le sujet de l'énergie stabilise également notre compétitivité à court terme mais aussi à long terme la loi une flèche nourri d'Action Act des États-Unis dont l'objectif est de boosté l'industrie verte et le secteur de la santé mettent en danger notre marché comment bien que l'objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 soit louable. Nous ne pouvons pas laisser partir nos industries. Nous ne pouvons pas voir notre marché commun envahis par des produits moins chers fabriqués hors Union européenne. Les règles de concurrence doivent rester équitable il faut stimuler et soutenir notre compétitivité, notre souveraineté n'est pas une option seuls notre indépendance doit nous guider. Le plan industriel vers présenté demain sera l'un des sujets majeurs de la semaine prochaine. La Commission européenne travaille sur la simplification d'accès aux financements aux aides d'État tout comme sur la facilité en matière de réglementation. L'objectif étant une transition juste et efficace cependant Madame la Ministre, pouvez-vous déjà nous indiquer. Les actions qui pourrait que pourrait mettre à Oeuvres le gouvernement afin que ces règles puisse s'appliquer rapidement et correctement sur nos territoires. Est-ce qu'une ingénierie local est prévue afin d'aider nos entreprises et nous citoyens qui font face aux complexités européenne et qui parfois se sentent bien démunis même s'il ne sera pas forcément à l'ordre du jour du Conseil européen. Notre relation avec le Royaume Uni. Nous avons longuement débattu de ce point dans cet hémicycle, nous nous sommes émus du choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Nous avons exprimé notre colère et nos craintes face à leur attitude lors des négociations de l'accord de retrait ainsi qu'après nous sommes restés ferme face au Northern Ireland protocole Bill et aux remous provoqués sur le sujet de la pêche. Nous avons tenté de formuler des solutions nous sommes restés suspendus bien des fois au vote du Parlement britannique et quelques fois à son refus. 3 ans après leur départ la relation semble enfin apaisé, tout, tout du moins les discussions le 27 février, le cadre de Windsor était est venue poser une nouvelle Pierre à notre relation nouvelle. Certains ont évoqué une normalisation. Nous partageons une histoire commune. Des valeurs communes, une vision commune sur bien des plans. Nous vivons sur le même territoire la relation Royaume-Uni Union européenne sera toujours au delà de la normalité car extraordinaire cependant Madame la Ministre. Est-ce que les règles négociées sur le statut de l'Irlande du Nord assure la protection du marché unique. Ma question se situe sur le volet pratique, sommes-nous sûrs de pouvoir matériellement assurer les contrôles et la coopération nécessaire en matière d'effectifs et d'infrastructures. Si ce n'est pas le cas à quel horizon. Serons-nous prêts plus largement. Pouvez-vous revenir sur les étapes qu'il reste ce pour entériner concrètement ce cadre. Le Conseil européen qui arrive étant encore une fois crucial. Comme à chaque fois, vous n'avez d'autre choix que de réussir. Mais vous avez aussi toute notre confiance. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Jacques Fernique du groupe écologiste pour six minutes. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le rapporteur général monsieur le vice-président monsieur le vice-président de la commission des affaires européennes. Effectivement c'est hier que la Commission européenne a présenté sa proposition de réforme du marché de l'électricité pour soulager les consommateurs en agissant sur les prix orienter le marché vers les énergies renouvelables et dépendre moins des coûts des fossiles. Alors que cette présentation ouvre une phase qui sera déterminante. Je pose nettement la question. Est-ce que, sur ces enjeux européens majeurs. Nous devons nous résigner à voir notre pays se comporter comme un petit pays de la négociation européenne obnubilé par la défense partout et toujours et tout le temps de sa spécificité nucléaire ainsi notre gouvernement s'est montré très actif pour développer les contrats à long terme, notamment pour soutenir le le nucléaire. On a obtenu pour faire plaisir à la France, l'Espagne propose donc de promouvoir les contrats différence pour les technologies qui ne sont pas soumises à la concurrence d'une nouvelle entrée sur le marché comme le nucléaire, ce lobbying s'étend a bien d'autres dossiers comme la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments par exemple ou les pressions pour inclure des objectifs de déploiement de l'hydrogène nucléaire dans le cadre réglementaire en cours de révision. Et pendant ce temps, la France est le seul État membre à devoir débourser 500 millions d'euros pour n'avoir pas atteint son objectif d'énergies renouvelables pour 2020. Seuls pays européens à la traîne autant pour l'éolien que pour le solaire. Électricité solaire dont dont le boom mondial et les bas coûts sont à présent avérés, la France persiste et signe dans la voie du nucléaire. Mais ce choix n'aura aucune utilité pour les 15 ans à venir. Le GIEC le martèle pourtant c'est dans les 10 ans que les principaux investissements de transition énergétique doit produire leurs résultats pour le climat. Chaque euro dépensé au profit d'un nouvel essor nucléaire sera, ce sera autant en moins pour le déploiement des renouvelables. La découverte de fissures pas négligeable du tout sur des réacteurs à Penly à quatre nomme les sécheresses plus fréquentes et plus marqué qui fragiliserait les localisations le long des fleuves, les déchets, les incertitudes sur un sur un financement absolument pas maîtrisé et un coût moyen de production d'électricité nettement plus coûteux. Autant d'arguments pour ne pas tout. Ainsi dans cette voie et dans un tel lobbying européen. Ce lobbying. Il est même cynique, ignorant la demande du Parlement européen d'un embargo immédiat notamment sur l'uranium russe. La commission a plié face au président Emmanuel Macron, elle a renoncé à l'instar du Conseil à sanctionner des cadres importants du nucléaire russe comme ceux de Rosatom entreprise créée par Poutine lui-même le nucléaire est à l'abri des sanctions en pleine guerre russe contre l'Ukraine, la France a quasiment triplé ses importations d'uranium enrichi provenant de l'aire d'influence russe et a exporté en 2022 vers la Russie l'intégralité de son uranium de retraitement. La France ne brille pas non plus par son exemplarité concernant la protection des océans. C'était la semaine dernière, notre secrétaire d'État à la mer ici même qui. Réussissent à l'exploit de qualifier le traité sur la haute mer d'historique, tout en défendant dans la même phrase bec et ongles le chalutage de fond dans les aires marines protégées. Quel est le sens de la notion d'aires marines protégées, si un ministre il défend des engins de pêche qui ravage les fonds marins des pratiques si destructrice de la biodiversité, l'écart entre les opérations de communication du gouvernement et ce qu'il défend réellement est sidérant. C'est pas moi c'est Jacques Attali qui s'en offusquent sur Twitter. Il serait grand temps d'écouter les scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer et de fermer les zones de pêche concernées pendant les pics d'échouage de dauphins tout en compensant financièrement les pêcheurs l'inaction du gouvernement en la matière. Entraîne la mort de plusieurs centaines de dauphins par an sur la côte Atlantique et lui vaudra sans doute bientôt d'être condamnée par la Cour de justice de l'eau de l'Union. À contrario de mes critiques sur les renouvelables et la protection des des biodiversité marine, je tiens à saluer le cap maintenu par le gouvernement concernant l'échéance européenne de fin de ventes de véhicules neufs à moteur thermique en 2035 le revirement allemand et sa tentative de monter une minorité de blocage est inacceptable. Comment le Parti libéral démocrate en déconfiture électorale de mèche. Il faut le dire avec des intérêts privés de petits et moyens constructeurs sous-traitants pourrait-il saboter les chances de nos constructeurs de répondre au défi chinois. Comment on pourrait le faire en contrecarrant ainsi l'échéance 2035 qui est une nécessité écologique et. C'est précisément le Green Deal et une stratégie industrielle qui ne soit pas très courte vue qui réduira l'écart avec les constructeurs chinois et contribuera à une réponse à la hauteur de l'IRA, ne laissons pas détricoter Green Deal, Ne laissons pas tuer dans l'oeuf les discussions sur la norme euro 7 qui viennent, il faut le dire très mal de démarrer tenons bon sur 2035. Enfin je salue aujourd'hui le vote au Parlement européen d'un revenu minimum européen. Il est temps de concrétiser l'un des objectifs affichés par l'Union qui est de réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2030 sur le continent et cela passe aussi par la jeunesse en France, une personne pauvre sur deux à moins de 30 ans, cette dynamique européenne dont témoigne le vote d'aujourd'hui ainsi que la France hein. Mettre un terme à la discrimination des moins de 25 ans dans l'accès au RSA. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein Monsieur André Gattolin du groupe RDPI et vous avez 9 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. L'Union européenne se trouve aujourd'hui dans une situation que je qualifierai des plus paradoxal, ce n'est pas la première fois de son histoire mais dans le contexte actuel extrêmement grave de la guerre en Ukraine ce paradoxe interroge et d'une certaine manière inquiète. En effet, après avoir honorablement fait face à 3 crises inédite qui aurait pu lui coûter son existence où la mettre en péril l'Union Européenne semble aujourd'hui potentiellement menacés par un banal accident de voiture. Alors je vous l'accorde. Mon propos sibyllins et un peu mystérieux mérite explication. Des trois crises que j'évoque ces trois crise inédite Sussex su successives. Ces 3 astre noirs qui ont fait l'un après l'autre irruption dans la paisible Galaxy Europe nous les connaissons tous la première crise est évidemment celle qui a résulté du Brexit. Pour la première fois de son histoire union a vu un de ses membres, et non des moindres claqué la porte en posant pour sa sortie des conditions parfois a saisi réaliste et la négociation fut longue et pénible et l'accord une fois trouvé fait encore l'objet de renégociation. Les divisions fratricides souvent prédite entre les 27 membres restants de l'Union n'ont cependant pas eu lieu et nous semblons même aujourd'hui. Apercevoir le bout du tunnel après l'accord de Windsor a évoqué par ma collègue collecte mélo entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui revisite, en des termes acceptables les pin-up protocole douanier concernant l'Irlande du Nord. Le sommet franco-britannique qui s'est tenu il y a quelques jours à l'Élysée vient également scellé les bases d'une nouvelle relation relation constructive entre nos 2 pays bien sûr et même si une proportion croissante de Britanniques dit regretter le choix du Brexit. Le Royaume-Uni n'est pas près de revenir sur sa décision historique. On note cependant que la nouvelle donne internationale et plus encore la dégradation de la situation économique outre-Manche semble ouvrir la voie à des relations plus apaisées et surtout à des coopérations accrues entre l'archipel et l'Union européenne. Alors Madame la Ministre pourriez-vous nous faire un point sur les perspectives précisément qui s'ouvre aujourd'hui à ce sujet. La seconde crise inédite. Ce fut celle de la pandémie de Covid-19. À la fois, sanitaire, économique et social, là encore, l'Union a assez vite réagi, notamment dans un domaine de la santé qui ne relevait pourtant pas de ses compétences propres. Elle a su réagir économiquement aussi avec un plan de relance sans précédent et une suspension des sacro-saintes règles sur le déficit budgétaire et l'endettement public autorisé. Après une récession très marquée en 2020 les économies européennes ont connu un robot rebond presque inespéré en 2021. Certes, tout ceci s'est fait au prix d'un endettement accru des États et la Commission appelle depuis quelques mois un retour au respect des règles budgétaires édictées par les traités européens. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelle est aujourd'hui la philosophie de la commission en la matière, notamment au regard des nouvelles conséquences lourdes notamment budgétaires qui résulte de l'actuelle guerre en Ukraine. Jean vient naturellement à la 3ème crise inédite affronter par l'Union, celle de la terrible guerre d'agression menée par la Russie depuis plus d'un an à l'encontre de l'Ukraine, avec son cortège déjà long de conséquences lourdes, tant économiques que politiques chronologiquement. Il s'agit de la plus récente des crises que je viens de lister mais rien malheureusement ne nous assure qu'il s'agisse de la dernière compte tenu de l'instabilité géopolitique globale qui règne désormais les soubresauts qui agitent le monde bancaire et financier ou de possibles nouvelles crise migratoire qui se profile. Notons également que même si ces trois crises paraissent se succéder dans le temps il est clair que certaines conséquences long cours des 2 premières viennent en partie se superposer sur l'instant présent le tout impactant simultanément nos économies et les équilibres politiques qui jusque-là s'imposait au sein de l'Union. Cependant, Cependant, et bien sûr avec toute la prudence qui sciait lorsqu'on s'aventure sur les Terres incertaine de l'avenir. Le 1er constat que l'on peut faire c'est que les l'union a réagi avec plus de rapidité et plus d'ampleur que nous n'aurions jamais osé l'imaginer avant la guerre, souvent qualifiée de réveil géopolitique de l'Europe et d'ailleurs il faut bien l'avouer, moins significative. On va l'oral hâtive qu'en volume des engagements pris. Nous frappe surtout en comparaison avec l'inanité qui prévalait dans la partie occidentale de l'Europe face à la menace extérieure. En valeur relative en comparaison avec les autres. Force est de constater que si progrès Elia. En revanche, on n'observe pas encore de ce qu'on appelle l'effet wahou qui ferait de l'Europe et qui la ferait entrer dans le cercle restreint des acteurs géostratégique qui pèse le plus dans notre monde en pleine recomposition. Pourtant il faut admettre qu'en dépit de la grande diversité des nations qui composent l'Union cette dernière là encore a fait preuve d'une grande et cohérence et résilience depuis le début du conflit. Alors bien sûr le cas de la Hongrie fait singulièrement tache dans ce tableau européen plutôt harmonieux Madame la Ministre, pensez-vous que monsieur Viktor Orbán puisse être en mesure de refuser et de bloquer d'éventuelles nouvelles mesures européennes en faveur de l'Ukraine ou contre la Russie et les deux mesures permettant l'adhésion future et et rapide de l'Ukraine à cette même Union. Notons qu'il existe au moins une conséquence positive qui résulte de l'attitude négative de la Hongrie, c'est celle d'avoir définitivement fait voler en morceaux et en éclats le fameux groupe de Visegrad qui a souvent en entraver la dynamique européenne au cours des 15 dernières années. Il faut se féliciter également je crois du rééquilibrage Est-Ouest qui semble ce pourrait s'opérer aujourd'hui à la faveur des événements au sein de l'Union le poids nouveau qui est pris par la Pologne et aussi la Roumanie pourrait favoriser à terme une meilleure intégration politique de ces pays dans une Europe qui n'a désormais pas d'autre choix que de se repenser. Plus généralement, et en dépit des réactions positives aux crises des dernières années. Nous restons dans les faits, encore loin de l'Union invoqué en guise de prophétie. Autoréalisatrice lorsque nous avons formellement décidé en 1993 d'adopter la dénomination d'Union européenne et objectivement et près de 20 ans après le grand élargissement, nous commençons à peine à nous commuée en une véritable communauté de nations et de peuples alors restons lucides. D'autant que le processus d'intégration à l'instar du processus démocratique n'est ni constant ni linéaire. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une régression et pour illustrer ce risque éclairer mon propos préalable sur un possible banal accident d'automobile qui pourrait mettre à mal l'Europe dans son fonctionnement je veux rapidement ici évoqué comme mon prédécesseur. Jacques Fernique l'attitude récente de l'Allemagne remettant soudainement hein, cause l'accord trouvé à l'issue d'un trilogue pourtant concluant sur la proposition de règlement, mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique à l'horizon 2035. Nous connaissons bien sûr tous l'importance de l'industrie automobile dans l'économie et même dans la politique allemande et nous sommes nombreux à nous rappeler l'empressement de Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission à se rendre à Washington en juillet 2018 pour tenter de convaincre le président Trump d'épargner une hausse de taxes d'importation aux véhicules européens comme par hasard à 80% allemand au détriment des alcools et des produits de luxe, comme par hasard essentiellement français et italiens. Alors je le dis ce type d'attitude est totalement délétère pour une juste et un juste et équitable fonctionnement interne de l'Union le cavalier seul qui fut par le passé opéré par l'Allemagne en matière d'de dépendance gazière excessive à l'égard de la Russie continue aujourd'hui de nous coûter collectivement très cher ici et ailleurs, nous avons tous salué la décision allemande d'investir enfin très significativement dans sa défense et dans la défense européenne très récente décision Berlin semble renouer avec une conception plus nationale qu'européenne plus mercantile que politique, de sa place au sein de l'Union, c'est une horreur je crois Madame la Ministre qui va convenir de corriger très vite, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jean-Yves Le compte du groupe socialiste pour cette minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. 55 milliards d'euros de. Recettes. De commerce en 2021, 431 milliards d'euros de déficit commercial en 2022. Voilà l'évolution de l'Union européenne. Une illustration de plus du choc et finalement de la remise en cause du volume de la remise en cause de notre modèle européen face à cela, je crois qu'il est indispensable de faire preuve d'humilité dans cette remise en cause mais aussi de solidarité. Car finalement tout le monde est responsable et chercher des boucs émissaires parmi nos partenaires ne nous permettrait pas de trouver en solidarité une réponse à ce qui est un défi commun trouver un un nouveau modèle sans se battre sur les questions de d'hydrogène de nucléaire de manière de produire l'hydrogène de manière de les transmettre. Nous devons plus que jamais et de manière encore plus résolu compte tenu de ce que nous avons vécu en 2022. Avancer vers le Green Deal. En solidarité et en sachant que nous trouverons ensemble une solution, cette solution ne la trouverons aussi ensemble parce que. Malgré tout les. les. Échos pessimiste que nous avons, nous sommes encore. Un espace fort en matière commerciale et cette puissance commerciale de l'Union européenne dans son ensemble. C'est un atout. Ce n'est pas un atout suffisant. Nous avons vu que si on fait du commerce sans s'aimer. Eh bien il y a le Brexit. Et que si on fait du commerce sans se comprendre. Et ben il y a un moment d'un choc et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec la Russie. Alors bien entendu. Chercher à construire. Des, un, un nouveau modèle passe aussi par la manière parce qu'il ne faut pas le construire en autarcie par des accords commerciaux mais des accords commerciaux qui sont des accords commerciaux qui sont assumées assumée par l'ensemble des populations

Quand nous entendons que la Commission européenne pourrait dissocier des accords commerciaux entre la partie strict. Strictement commercial, comme on l'entendait dans les années 80 et la partie plus politique pour éviter de passer devant les Parlements, les parlements nationaux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas correct, si nous avons des bons accords politiques et des bons accords commerciaux. Alors nous pourrons avancer, mais en tout état de cause, faire des accords commerciaux comme au siècle dernier n'est certainement pas la manière de placer l'Union européenne en position de force et tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent sur nos faiblesses par rapport à, à des questions comme les aides d'État mérite aujourd'hui que nous construisions les choses de manière différente, plus politique et que la, la Commission européenne sache avancer avec l'ensemble des parlements nationaux. Et que nous ne nous trouvions pas devant défaite accompli en matière d'accords commerciaux. Vis-à-vis. De la situation en Ukraine. Nous devons plus que jamais nous mobiliser pour être aux côtés de l'Ukraine où lui faut dire les armes qui lui permette demain d'être en situation d'imposer la paix sur son territoire d'être aux côtés aussi des réfugiés que nous accueillons de faire en sorte aussi que nous reconnaissions le fait que la CPI doit pouvoir lancer des mandats d'arrêt contre toutes les personnes responsables de crimes de guerre en Ukraine et je dois saluer de ce point de vue-là, ce qui a pu être fait. Pas André Gattolin sur la proposition de résolution européenne relatif aux aux enfants toute la chaîne de commandement, des écussons de ce qui peut être qualifiée comme un Crime de génocide ne doit. Faire ne doit avoir aucune impunité. L'État de droit. Doit être aussi plus résolument que jamais défendu, nous le devons au peuple ukrainien à ses souffrances et à son combat. Résolu auprès des pays membres. Et aussi auprès des candidats à l'Union européenne Ukraine en 1er lieu l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, la liberté de la presse cette opinion. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Nulle part dans l'Union européenne est nulle part parmi les candidats. Ce que nous avons fait en donnant. À l'Ukraine, la qualité de candidat à l'Union européenne est une bonne chose. C'était indispensable mais ça doit maintenant être. La source d'un nouveau dynamisme pour l'ensemble des pays candidats, en particulier des pays des Balkans qui ne croit plus à cette perspective européenne et nous devons trouver pour demain des nouveaux dynamisme pour crédibiliser cette. À cette perspective d'adhésion qui. Mérite d'être crédibiliser pour les pays les peuples des Balkans

d'AD et d'avancer. Ce qui a pu être fait, il y a quelques années en matière de de véto vis-à-vis de la Macédoine doit faire partie du passé, il faut trouver un nouveau dynamisme pour. Les perspectives d'adhésion, même si elles seront difficiles. Bien entendu, ce sera difficile de l'Ukraine et est une puissance agricole comme il y en a probablement pas d'autre. Sur l'ensemble du continent et ce sera difficile mais il faudra avancer et ça sera bon pour l'ensemble des pays européens. Enfin en conclusion je voudrais aussi dire qu'il est indispensable sur les questions du pacte Migration d'avancer, pas simplement sur Eurodac, pas simplement sur le screening, pas simplement sur ce qui est entre guillemets répressif mais sur les aspects de solidarité et en prenant totalement en compte. les enseignements de ce que nous avons pu faire avec la protection temporaire, c'est-à-dire avec la liberté de circulation dans l'ensemble de l'Union européenne et le droit au travail pour les personnes que nous avons protégé et qui venait d'Ukraine. en conclusion Madame la Ministre permettez-moi de sans évoquer l'ensemble des relations entre l'Union européenne et l'Afrique et sa politique de visas qui me semble être particulièrement préoccupante dans la manière dont. Notre. Europe et notre pays sont perçus aujourd'hui en Afrique. Je voulais simplement faire partager mon inquiétude sur l'évolution de la Tunisie. L'Europe ne peut pas être tétanisé face à un pays dont probablement l'avenir et dans la relation avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. En imaginant simplement le pire pour ce pays avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir l'Europe. N'est jamais vraiment elles-mêmes que lorsque elle est fidèle à ses valeurs et qu'elle se tient tout en étant conscient de son histoire et qu'elle se tient résolu aux côtés de la liberté de l'ensemble des peuples du monde. Cela vaut pour l'Ukraine. Cela vaut pour l'ensemble des peuples du monde et lorsque nous savons dire avec les peuples qui réclament la liberté. Femme, vie, liberté, comme c'est aujourd'hui le combat du peuple iranien dont nous devons aussi être solidaire et l'Union européenne aussi doit marquer sa solidarité sans. Limite avec ses combats. C'est ainsi et c'est pour cela que l'Union européenne doit être plus forte et doit se développer.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans cette période de disette de progrès social. Je vais commencer par me réjouir. Oui, je vois que le Parlement européen a entériné avec 376 votes pour son adoption la directive consacrant la présomption de salariat des travailleurs des plateformes. Avant un débat tronqué. Sur les retraites, Emmanuel Macron aurait dû présenter au préalable une loi sur le travail. Dans ce texte, la France serait honorée à reconnaître le salariat des travailleurs des plateformes avant même la fin du processus législatif européen. Pourtant le président Macron en a décidé autrement. La réforme des retraites apparaît comme un solde de tout compte. Oh, mettant le débat primordial sur le travail, en particulier des travailleurs ubérisés qui cumule et les précarités et eux qui eux ne connaîtront pas les retraites. Par cet acte manqué, c'est quand même 6 milliards d'euros. Qui échappent aux caisses de la Sécurité sociale. Voilà une piste de financement du système des retraites 1,25 milliards pour les retraites. La dignité pour les travailleurs. C'est ce qu'on dirait une manière familière une pierre deux coups. super. Par les luttes et les décisions judiciaires le repas franchi une première étape malgré une évolution du rapport de force en faveur de la requis requalification des travailleurs et du droit du travail. Le président de la République reste arc-bouté sur une défense obstinée des intérêts des plateformes Madame la Ministre je vous le demande le gouvernement continuera-t-il d'être récalcitrants à cette avancée sociale. Mieux, prévoyez-vous de devancer l'adoption définitive de la directive pour consacrer dès demain un droit nouveau pour les travailleuses et les travailleurs des plateformes. S'agissant de la réforme des retraites, le contrat pourrait d'ici au 23 mars être remplies. La réforme des retraites ainsi adopté contre l'opinion populaire majoritaire. Nous ne cesserons de rappeler que comme pour l'Espagne. Cette réforme des retraites est exigée par la Commission européenne et il y a dans cette affirmation nul complotisme ou projet dissimulé tout est transparent. Tout est public et vous le savez madame la Ministre, le 5 juin 2019, le Conseil de l'Union européenne enjoignait la France à réformer les retraites, bis répétita. Le 1er juillet 2022. Les ministres des États membres de l'Union je cite recommande que la France attache en 2022 et 2023 à réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite afin de renforcer l'équité du système tout en soutenant sa durabilité, fin de citation. Vous nous direz peut-être pas ce soir, on a déjà eu beaucoup de temps de débat mais quelle équité dans cette réforme. La commission, tout comme le Conseil raffolaient d'une retraite par points, comme le prévoyait la précédente réforme mise en échec en 2019, elle préparait plus frontalement plus frontalement mais j'irai dire moins sournoisement l'accroissement d'une part de capitalisation. Le recul de l'âge de départ obligera ce qui le peuvent à mettre de côté pour se prémunir des des côtes de l'épuisement professionnel ou des minima sociaux et, cette manne va être captée par le système bancaire, puis placé sur les marchés financiers. D'ailleurs les banques américaines font faillite sans garantie des dépôts et sans garantie déplacements ça devrait quand même nous faire réfléchir et je vous le dis il suffit pas de crier calme donne comme Bruno Lemaire. Pour faire cesser l'irrationalité des marchés devenus fous la pression européenne pour une réforme des retraites, un phénomène de longue date en France comme en Europe en gouvernant par pression et en mettant des réformes contre le progrès social, je vous le dis avec solennité, Madame la Ministre on réarme les extrêmes droites dans leur quête du pouvoir. Le tout sur fond d'affaiblissement continu des parlements nationaux, et là on réunit les conditions d'un régime autoritaire. Je vous le dis aussi notre idéal démocratique et bien mise à l'épreuve. La contre-, réforme des retraites n'est pas la seule volonté d'ingérence de l'Union Européenne dans la souveraineté budgétaire des États après leur suspension pendant la crise sanitaire, les règles budgétaires reviennent et seront probablement abordée au point 3 de l'ordre du jour du conseil. Nous attendons les éléments mais ce que nous entendons est extrêmement préoccupant et ne rien les leçons des volontés austéritaire inapplicable et inappliquée 3% de déficit. Une hérésie. 60% de dette publique. Excusez-moi une fable répété à l'envi le peuple souverain a-t-il décidé de telles règles. Moi j'ai du mal à en trouver la traçabilité démocratique et alors je vous le dis bah pourquoi pas oser consulter les Parlements nationaux. Et en tout état de cause, la Commission a présenté le 9 novembre 2000 vide 2022 une nouvelle méthode. Chaque État pourra définir lui-même sa propre trajectoire de réduction des déficits et de sa dette publique, le tout sur 4 ans. Il serait terminé des règles uniformes qui n'ont jamais fonctionné. Mais si un délai supplémentaire de trois ans est prévu pour les pays dont la dette publique dépasse 60% du PIB. Ce serait et là je cite. À condition que les États membres s'engagent à adopter des réformes structurelles et à faire des investissements stratégiques de nature à alimenter la croissance. en gros, pour résumer réforme stricte Turrell mais quand même sous. Le patronage d'un chantage. Un chantage amener des contre-réformes libérales contre l'intérêt des classes populaires et on peut se poser la question peut-être vous nous donnerez dans les modes réponse quelle croissance. Une croissance pour qui. Pour quels nouveaux emplois pour quel nouveau métier pour quel progrès sociaux. Je crois qu'on ne peut pas raisonner seulement par la croissance pour la croissance. Il me semble que ça peut une impasse. J'ai pu regarder dans un média allemand qui régime ainsi les annonces de la commission, je le cite plus de marge de manoeuvre mais aussi plus de rigueur. J'ai du mal à voir les marges de Madoff. Mais je vous avoue Madame la Ministre je vois bien la rigueur. Maintien de la procédure d'infraction pour déficit excessif. Rien qu'à entendre l'expression c'est qu'on va prendre perpétuité et là sans remise de peine. Renforcement des sanctions relatives au niveau de la dette publique par des sanctions financières des sanctions de réputation notamment par une convocation à une audition au Parlement et blocage des fonds structurels. Et là, rassurez-vous, mais quelques collègues qui comme moi sont assidus à cette soirée. Le tout cela sera préventif bien évidemment le goulot d'étranglement interviendra plutôt en fermant les États dans l'austérité en asséchant leurs capacités budgétaires en gros les mêmes causes auront les mêmes effets et s'il faut prendre une référence au niveau de notre beau continent, l'Europe, je crois que la Grèce en a fait durement les frais. En plus ces deux piliers du pacte de stabilité sont maintenus. Déficit public limité à 3% du PIB, un plafond d'endettement à 60%. Parce que les finances publiques, ce n'est pas qu'une dette c'est aussi un Patrimoine financier et immobilier. Je vous le redis, là on a déjà l'occasion d'expliquer mais la dette de la France ne serait plus de 87% et non 115% si on procédé ainsi on nous roi penchant ainsi de l'objectif infondées de 60% nos concitoyens nos consulte ivoirienne aurait le droit de décider de leur propre politique. Voilà les éléments que je voulais livrer à votre réflexion. Merci de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Jean Michel Arnaud du groupe Union centriste et vous avez 7 minutes. Madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis concentrée principalement mon propos sur les volets relatifs à la compétitivité et à l'énergie inscrire lors du jour de la prochaine réunion du conseil. La crise énergétique a affecté la balance commerciale de la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Dont le déficit s'établit à 160 milliards d'euros en 2022 pour la France. Les subventions massives aux technologies vertes. De l'inflation réduction Act américain laisse craindre une nouvelle perte de compétitivité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Le 8 février dernier, le Sénat a ainsi consacré un débat d'actualité. À la question suivante. Quelle réponse européenne aux récentes mesures protectionnistes américaines. Madame la Ministre, comment éviter un détournement l'investissement européens vers les États-Unis. Faut-il ouvrir la voie à de nouveaux financements pour nos industries vertes ou miser sur le renforcement de l'enveloppe existante comme le Fonds européen développement régional Feder. Le renchérissement récent du dollar vis-à-vis de l'euro semble représenter une opportunité de relance pour la politique industrielle européenne. Dès lors qu'il est porteur de gain de productivité et de compétitivité. Pour nos entreprises exportatrices. Mais comment éviter une course aux subventions entre États membres qui fragiliserait les règles de concurrence équitable sur lequel est bâti le marché unique. La dégradation du solde notre balance commerciale. Procède principalement de la dépendance de l'Union européenne à l'égard des énergies fossiles. Il convient de prendre les mesures nécessaires au renforcement de la souveraineté énergétique du continent. Je salue le fait que depuis peu les plans nationaux de relance et de résilience peuvent compter un chapitre oui pour You qui leur permet d'accéder aux 20 milliards d'euros dans 2 milliards 320 millions pour la France de subventions supplémentaires prévus dans le cadre de ce plan européen. Je m'interroge toutefois sur la possibilité donnée aux États membres de puiser dans les fonds de réserve de la politique de cohésion à hauteur de 7,5% de fédère. Mes chers collègues, cela ne risque-t-il pas de priver nos régions de financement essentiels à leur développement économique, madame la Ministre des mécanismes de compensation du manque à gagner pour nos territoires sont-ils envisager. De manière générale, il est regrettable que les collectivités étaient tenus à l'égard de l'élaboration des plans de redressement et de résidence nationaux. Je note que ces plans doivent désormais contenir une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales mais comment garantir que leurs besoins sont réellement et seront réellement pris en compte dans le texte final. Par ailleurs, je souhaite vous interpeller sur la feuille de route qu'a présenté Kadri Simpson. Commissaire européenne, responsable de l'énergie hier devant le Parlement européen. 3 mesures majeures, on était à non été annoncés. La première, la réforme proposée maintient le système dit du mérite hors selon lequel la dernière unité de production électrique fixe les prix. L'exécutif européen n'a pas accédé à la demande française d'un découplage total entre le gaz et l'électricité. Deuxièmement, pour les nouveaux investissements dans le bas carbone là où un financement public est nécessaire. La commission plaide pour le recours à des contrats pour la pour la différence. Ce qui représenterait une opportunité pour nos investissements dans le nucléaire. Enfin la proposition oblige également les États membres à établir des fournisseurs en dernier ressort afin qu'aucun consommateur ne se retrouvent privés d'électricité mais vise aussi à renforcer la capacité de surveillance de l'agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie et des régulateurs nationaux. Madame la Ministre, quelle sera la position de la France dans les négociations à venir sur ce sujet particulièrement sensible à la fois pour les industries nos entreprises mais aussi pour les consommateurs. Un autre point que je souhaite souligner et le plan des mobilités. L'Allemagne vient de de surprendre tous ses partenaires européens et la France en particulier en s'opposant un texte européen censé imposer la vente de véhicules uniquement électrique à partir de 2035. Ce faisant, elle a entraîné dans son sillage plusieurs autres pays d'Europe centrale. La Hongrie en particulier mais pas que. Ou l'industrie automobile et puissante et représente une part importante de l'économie. Cette décision doit nous amener à réfléchir à des alternatives au tout électrique qui nous permettrait de nous détacher des énergies fossiles sans pour autant imposer une technologie précise aux industriels. Depuis quelques jours le gouvernement français est sollicité pour savoir quelle est sa position par rapport à cette proposition de Berlin. D'utiliser les carburants synthétiques dans les moteurs à combustion après 2035. Quelle voit la France entend-elle porter au conseil alors même que plusieurs de nos producteurs et constructeurs automobiles, comme Renault se sont engagés à fabriquer 100% de véhicules 0 émission en Europe dès 2030 et que Stellantis prend visiblement la même orientation tout en étant, en ayant été beaucoup plus critique que Renault sur ce sujet. L'actualité européenne sera également bientôt marquée par l'entrée en vigueur de de directives ayant pour objectif une meilleure régulation numérique. Pour rappel à eux seuls les Gafam représente un chiffre d'affaires comparable aux recettes fiscales de la totalité de nos leur modèle économique qui repose sur la combinaison de masse de données sur leur utilisateur et sur des algorithmes puissants et opaque leur permet d'avoir une position de quasi-monopole sur le marché européen, laissant peu de place à la concurrence. Cela appelle alors une nouvelle régulation européenne dans les prémices verront le jour avec les directives dites DMA et DSA. La DMA applicable au 2 mai 2023, vise à stimuler l'innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché numérique ainsi qu'à renforcer la liberté de choix des consommateurs européens en créant une concurrence loyale entre les acteurs du numérique. Quant au DSA applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche concernés dès 2023 il veut mettre en pratique le principe suivant, ce qui est illégal hors ligne et illégal en ligne. Il permet ainsi de s'assurer du bon fonctionnement du marché intérieur numérique avec des règles uniformiser. Quelle sera la position Madame la Ministre de la France au sein du Conseil européen pour favoriser effectivement ce travail et atténuer autant que possible des risques systémiques tels que nous avons pu constater, notamment à l'occasion du Brexit mais pas que. Mais également lors de grandes échéances électorales dans des pays de l'Union européenne, et bien au-delà, telle que la manipulation de l'information ou la désinformation. Je crois effectivement que c'est un sujet important pour nos concitoyens. C'est ainsi est important également pour donner démocratie et pour l'équilibre de nos démocraties, en Europe, attaqué à la fois et une enquête une mission d'information est lancé sur TikTok ici dans cette assemblée par des puissances extérieures mais aussi des manipulations à grande échelle qui font que, en Europe la question démocratique peut être aussi remis en cause par un manque de volontarisme en la matière j'attends effectivement de la part du gouvernement français et du Conseil de l'Europe des avancées sur ce sujet protecteur des libertés individuelles et de nos démocraties locales merci. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Martine Berthet du groupe Les Républicains et vous avez 8 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Guerre en Ukraine. Difficultés d'approvisionnement en matières premières et pénurie de semi-conducteurs, inflation et hausse sans précédent des prix de l'énergie, l'Europe traverse une grave période de turbulences. Le doublement voire le triplement ou plus des factures d'électricité et de gaz. Mais nos collectivités et nos entreprises dans une situation financière délicate. De sérieuses menaces planent sur la vie économique de nos territoires et nous le savons tous, l'indemnisation des collectivités et des entreprises par l'État ne peut durer car elle ne fait qu'aggraver plus encore notre déficit public quant au bouclier tarifaire il protège nos menace de la violente inflation des prix de l'énergie mais pour combien de temps. Dans ce contexte si un constat doit faire l'unanimité, c'est bien celui de l'incapacité du marché européen de l'électricité à protéger les consommateurs de la crise liée à l'approvisionnement en gaz. Cet aveu d'échec. La commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simpson l'a reconnu, le 27 février dernier à l'issue d'une réunion informelle des 27 Ministre de l'énergie de l'Union Européenne aujourd'hui les Français ménages entreprises TPE-PME industrie collectivités pâtissent de règles européennes dépassé qui font dépendre de façon paradoxale, le prix de l'électricité du cours des énergies fossiles que sont le gaz ou le charbon, alors même que notre pays produit une électricité peuchère grâce à son parc nucléaire et à son hydroélectricité. Nous ne pouvons sacrifier notre tissu économique et social Madame la Ministre mettre le pays tout entier en danger pour conserver quoi qu'il en coûte un marché européen de l'électricité dérégulé, qui ne joue plus son rôle. Le mécanisme ibérique qui consiste à intervenir sur le marché pour faire baisser les prix mis en oeuvre par nos voisins portugais et espagnols en témoigne. Il est efficace pour ces deux pays, mais il génère une concurrence déloyale pour nos entreprises. La réponse à la crise énergétique doit être une réponse commune aux membres de l'Union. Nous avons été nombreux à alerter le gouvernement sur ces différents écueils lors de sa déclaration de politique énergétique devant le Sénat le 12 octobre dernier. Madame, la Première ministre avait elle-même reconnu la nécessité de réviser les règles européennes. Pourtant, à la lecture du paquet législatif annoncé par le Madame Simpson hier au Parlement européen, la Commission européenne ne semble pas prendre la mesure des dysfonctionnements. Si l'objectif affiché de ces propositions. À ce que l'énergie produite sur le continent européen n'est pas un prix trop volatile et dépendants de nos importations de gaz et de pétrole si si cet objectif est tout à fait louable, il ne renvoie cependant qu'à des mesures ciblées, suggérant ainsi qu'aucune refonte refonte complète des règles n'est véritablement. Le système du mérite Order selon lequel la dernière unité de production électrique appelé fixe le prix est ainsi conservée et le découplage du prix du gaz de celui de l'électricité que nous appelions de nos voeux n'est toujours pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, la Commission européenne a présenté des propositions sur l'industrie zéro carbone. Elle souhaite lancer une stratégie de décarbonation massive de nos productions industrielles qui inclura toutes les modalités d'une production énergétique neutre en carbone. Or sur ce point, la commission est revenue sur sa proposition initiale en excluant le nucléaire du domaine des énergies qui doivent pouvoir être utilisées par une Europe qui se décarbone. Dans la perspective d'une réforme du marché européen de l'électricité c'est un anachronisme pour rompre avec des logiques de production polluante et carbonée. Il faut nécessairement faire avec le nucléaire. Le GIEC nous le rappelle régulièrement. Les traités européens garantissent. Aux États membres le droit et le devoir de définir souverainement leurs propres mix énergétique. L'Union européenne doit simplement leur en donner les moyens. L'Allemagne dans le même temps double sa production de centrales à gaz, énergie fossile, faut-il le rappeler et place l'Europe dans une situation de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ce n'est pas acceptable. La France doit se faire entendre. Le nucléaire fait partout son retour au Moyen-Orient au Japon, en Chine, en Inde, au Canada, aux États-Unis, comme le rappelle Monsieur Fathi Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, l'Europe ne doit pas manquer ce saut technologique. Face aux stratégies de concurrence agressive et protectionniste auquel se livrent plusieurs de nos partenaires commerciaux depuis quelques mois la stratégie française lors du prochain conseil doit être sans ambiguïté aucune, la réforme du marché de l'électricité est un véritable enjeu de souveraineté économique et de compétitivité. Nos entreprises subissent en effet une double peine infligée par les États-Unis avec l'inflation réduction Act et par l'absence des choix européens fort et structurant. Ceux-ci sont pourtant essentiel pour que d'une part nous puissions profiter pleinement des avantages comparatifs que nous procure le nucléaire, énergie bas-carbone et que d'autre part l'indépendance économique européenne sorte renforcés de ce temps de crise. La réforme du marché de l'électricité doit pouvoir inciter des industriels européens et français aux relocalisations et nous permettent d'accélérer les investissements de transition vers une économie décarbonée et moins dépendante des économies étrangères actuellement la situation de notre industrie est préoccupante, elle n'a aucune visibilité sur ses coûts d'approvisionnement en électricité. À l'inverse, ses concurrents au niveau mondial disposent eux d'une visibilité de 10 15, 20 ans au minimum et peuvent se fournir en électricité à bas autant qu'il le souhaite. Pour ces entreprises l'électricité peuchère et parfois l'élément de base de leur production qui leur permet d'être compétitive vis-à-vis de leurs concurrents. À cet égard le rétablissement des contrats de long terme est indispensable pour sécuriser des prix d'approvisionnement stable et des coûts de production compétitifs. Mon département de la Savoie compte plusieurs grandes industries hyper électro-intensives qui produisent des matériaux nécessaires à la transition énergétique. Si ces entreprises ne peuvent renouveler leurs contrats de long terme en 2023, elles seront contraintes de baisser voire d'arrêter leur production. Certaines l'ont déjà fait en ce début d'année. La seule alternative est ensuite la Chine ou la Russie. Le déficit de notre commerce extérieur et la situation géopolitique de notre pays s'en trouverait aggravée. Le rétablissement de ces contrats fait partie des mesures ciblées par la Commission européenne. C'est une excellente nouvelle. Mais il faudra veiller à ce que l'adaptation du marché de l'électricité à un système énergétique dominée par les énergies renouvelables souhaitée par la Commission prenne bien en compte la production nucléaire afin de ne pas pénaliser nos industries dans la renégociation de leur contrat. La reconnaissance de l'urgence d'une nouvelle politique énergétique pour accélérer la décarbonation de l'économie et renforcer la compétitivité des entreprises européennes fait l'unanimité. Saisissons donc l'opportunité de ce prochain conseil européen pour défendre une réforme plus ambitieuse du marché de l'électricité. L'heure n'est plus aux déclarations d'intentions mais aux actes forts. La France doit se faire entendre. Le sujet d'ailleurs des concessions de nos barrages hydroélectriques n'est toujours pas réglé. Le gouvernement doit défendre nos intérêts Madame la Ministre nous comptons sur votre action. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein. Monsieur Patrice Joly du groupe socialiste pour 7 minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, en l'espace d'un an le paysage énergétique a considérablement changé. Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de 100%, ceux du charbon de 400% et les prix du gaz européen jusqu'à 1000%. La hausse des prix de l'énergie à alimenter la crise du coût de la vie qui touche d'autant. Plus Plus les foyers européens que leurs revenus sont modestes à l'impact aussi fortement les entreprises en particulier les PME et les TPE. Voilà. Jusqu'à présent, les États membres ont majoritairement réagit en instaurant des mécanismes d'urgence de contrôle des prix ou d'amortisseurs. Baisse de la fiscalité bonus climatique chaque énergétique ou chèque de chauffage. Alors que les prix de l'énergie sont loin d'être stabilisée. La réforme ciblée du marché de l'électricité proposée hier par la Commission européenne est-elle suffisante. Nous pouvons partager l'essentiel des objectifs affichés par la Commission, c'est-à-dire un accès généralisé et à un prix abordable. À l'électricité produite à partir des sources renouvelables et non fossiles. Une meilleure transparence des informations sur les marchés vis-à-vis des consommateurs. Et un plus grand choix de fournisseurs afin on consommateur de se trouvent privés d'électricité. Un accès amélioré des entreprises à des contrats et à des marchés. Ah le long terme plus stable, une révision des règles relatives à la revente des énergies renouvelables. Cependant, cette réforme ne devrait pas toucher aux fondamentaux. Du fonctionnement du marché alors que l'explosion historique des prix de l'énergie que nous subissons aujourd'hui en Europe. Provins provient bien de la défaillance du marché. De plus, le découplage strict gaz électricité. N'est pas prévu. Comment expliquer cet échec dans la négociation, alors que le ministre de l'économie en faisait son principal cheval de bataille. Ensuite nous ne maîtrisons pas le calendrier de mise en oeuvre. Le Parlement européen, le Conseil doivent désormais discuter et adopter cette proposition. Enfin certains experts et professionnels du secteur ne sont pas sûrs que les mesures présentées par la Commission flash pardon refluer les prix. La baisse des prix dépendant de beaucoup d'autres facteurs comme, La disponibilité du nucléaire français. La météo, le marché mondial du gaz notamment. Se pose alors plusieurs questions. Comment les ménages vont-ils passer l'hiver prochain. Les ménages verront-ils pour autant leur pouvoir d'achat préserver. Les entreprises bénéficieront. Attends d'une énergie à tarif compétitif. Au risque dans le cas contraire d'une course aux délocalisations. Au moment où les États-Unis renoue avec le protectionnisme pour protéger relocaliser et investir dans l'industrie verte, le coût de l'énergie coup fondamental au sein des coûts de production est aussi le nerf de la guerre. Car que penser de ce texte qui se présente aussi comme l'une des facettes de la réponse européenne à loi de réduction de l'inflation. Dite IRAM soit le plan américain de soutien massif à l'économie, qui comprend notamment de fortes. Subventions à l'énergie pour en baisser le prix. L'Europe veut-elle s'aligner pour ne pas dire que l'Europe doit s'aligner, car de nombreux défis de taille sont menées, dont ceux de la reconquête industrielle et de la transition écologique, qui ne peuvent plus attendre. Ce plan massif d'aide à la transition énergétique lancée par Joe Biden a montré à quel point l'Union Européenne est fondée sur un logiciel pseudo-économiques qui arrive à son terme. L'IRA ne doit pas se résumer en une tentative protectionniste américaine pour attirer l'industrie verte, en plein essor sur son territoire, au détriment de ses partenaires commerciaux. Joe Biden s'est engagé vendredi. Les derniers auprès d'Ursula von der Leyen à ne pas mettre en place une concurrence délétère dans la course à la transition énergétique et je le cite, travailler pour éviter une compétition à somme nulle afin que leur politique d'aide publique, soutiennent le développement des énergies propres. Et de l'emploi sans devenir des aubaines pour les intérêts privés. Fin de citation. C'est aussi une bonne nouvelle, de savoir que les États-Unis souhaitent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 même si on peut être dubitatif. À la suite de l'autorisation récente accordée pour l'exploitation du pétrole en Alaska. C'est aussi une belle opportunité pour l'Europe. Nous prenons collectivement conscience qu'il faut certes avoir une politique de défense vis-à-vis de la concurrence mais qu'il est vital de mettre en place une politique. Industriels et de transition écologique le jeu pour l'Europe se situe bien là, il s'agit d'accélérer les investissements bas-carbone dans le logement et la mobilité pour se préparer au prochain y va au prochain hiver en s'attaquant à la racine de la crise, à savoir notre dépendance aux combustibles fossiles. Il nous faut décarboner dès que possible, conformément au Pacte Vert la décarbonation et la. Et la compétitivité vont de Pair. De plus la transition ne peut se faire sans prendre en compte le pilier social. Nous ne pouvons pas parvenir à la durabilité environnementale 100 durabilité sociale. Il nous faut continuer à augmenter le budget du fonds social pour le climat. Sa portée pourrait contribuer à limiter la crise climatique. Et ce social et à garantir la sécurité énergétique tout en renforçant la solidarité européenne. Il est également essentiel que l'industrie soit préparé aux objectifs du Pacte Vert de neutralité climatique à échéance 2050. L'industrie de l'Union européenne doit avoir une position de leader international pour garantir notre autonomie stratégique et pour créer des emplois de qualité pour tous les Européens. Or pour faire de la politique industrielle et de la transition écologique. Il nous faut des subventions. Il nous faut de la planification, il nous faut des pouvoirs publics fort et il faut parfois aussi protéger nos industries. C'est pourquoi plusieurs leviers financiers doivent être activée notamment la. L'occasion de la revue à mi-parcours du cadre financier pluriannuel qui doit aussi avoir lieu d'ici l'été 2023, l'Union doit plus que jamais aujourd'hui se doter de nouvelles ressources propres à l'occasion m'a déjà été donné à de multiples reprises ici de dire combien il est important de disposer de moyens je pense bien sûr et vous y pensez également à l'extension des marchés carbone à la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone France tire le plus rapidement possible ou encore la création d'une nouvelle taxe sur les transactions financières et enfin une meilleure taxation des des bénéfices des multinationales. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent hein monsieur Olivier Cadic, à nouveau, mais là pour le groupe Union centriste et vous avez six minutes.

parler opportunisme opportunément des menaces que la Russie. Fait peser sur la Moldavie. De son côté la Géorgie fait face à un mouvement contestataire d'ampleur depuis le 7 mars dernier, date à laquelle le Parlement a adopté la loi dite des agents étrangers. Inspirée de la législation russe, le projet était censé museler les ONG et médias d'opposition dans le pays. Des rassemblements spontanés de plusieurs milliers de personnes à Tbilissi, la capitale ont fait plier le gouvernement. Quel avenir proche pour la Géorgie, pays paradoxal qui est dirigé par gouvernement inféodé à la Russie mais dont la population est acquise à plus de 80%. Ah la cause de l'Europe. En début de semaine. Sergueï Lavrov n'a pas hésité à comparer ce soulèvement à la révolution ukrainienne de 2014 dénonçant par là même des influences cherchant à provoquer un sentiment anti-russe. Et le représentant des affaires étrangères de la Crimée de de renchérir, nous recommandons peuple géorgien de se souvenir d'une situation similaire en Ukraine en 2014 et de ce à quoi elle a finalement mené. En juin dernier, l'Union européenne ces décrets re-prête à donner le statut de pays candidat à la Géorgie. Quelles sont les prochaines étapes envisagée sur cette adhésion les priorités nécessaires l'activation de ce statut sont-elles réunies. La situation de la Géorgie fera-t-elle l'objet d'un point précis lors du Conseil européen de la semaine prochaine. à libérer les stocks de munitions déjà existants. Il a passé de nouveaux contrats. Comme l'a mentionné le président Rapin, Thierry Breton a des. Tailler cet enjeu est existentiel pour l'Europe en expliquant qu'il fallait identifier les goulets d'étranglement qui empêche l'Union européenne de produire des munitions de manière massive et de faire avec les entreprises qui produisent de munitions presque du cas par cas cette stratégie permettra-t-elle à court terme de produire plus de munitions et de préserver notre souveraineté européenne sur le sujet. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur la proposition de résolution de mon collègue André Catelin déjà évoqués par notre collègue. Colette Mélot. Voter il y a quelques jours par la commission des affaires européennes. Elle sera examinée par la commission. Commission des Affaires étrangères et de la Défense dans les tout prochains jours. Elle dénonce des transferts forcés massives d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. La France et plus largement l'Union européenne. Mettront tels des moyens pour enquêter sur ces disparitions d'enfants. Enfin, je souhaite vous alerter sur le sujet de l'indopacifique. Le président chinois a apporté son appui politique à Moscou. Comme Poutine il combat le monde démocratique. Et cherche à le soumettre. Alors que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Affirment leur stratégie dans l'Indopacifique. Et en fait une déclaration commune. Il y a quelques jours l'Union Européenne peinent à fournir une réponse à la hauteur des enjeux de la région. En septembre 2021. Cette dernière a présenté sa stratégie pour la région indopacifique voulons répondre aux grands défis mondiaux en matière de sécurité, de climat ou encore de transition numérique. La zone est au centre d'une concurrence géopolitique très intensive. Preuve en sont notamment les tensions croissantes autour de territoire et de zone maritime contestée par la Chine, qui affiche son expansionnisme. La cheville Chine augmente encore. Son budget militaire investi dans sa capacité à prendre le contrôle de Taïwan et à exclure les États-Unis hors de la région. En décembre 2022, le Japon a modifié radicalement sa doctrine de défense. Et prévoit de doubler son budget annuel en le faisant passer d'environ 1% de son PIB à 2% d'ici à 2027 le mois dernier à Manille, le président Marcos a convoqué l'ambassadeur chinois pour dénoncer l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des actions menées par la Chine contre les garde-côtes philippins et ses pêcheurs. En février, les États-Unis et les Philippines ont signé un accord pour créer 4 bases militaires américaines supplémentaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Compte tenu de la proximité de Taïwan et de ses eaux voisines. Les Philippines occupe une position stratégique dans les vents actualité d'un conflit avec Pékin pronostiqué par certains généraux dès 2025. La situation dans l'indopacifique n'a jamais été aussi dangereuse depuis la 2ème Guerre mondiale nous a dit Julian Bird ambassadrice d'Australie en France. La France a toujours eu la volonté de porter une stratégie européenne sur ce sujet. Est-ce que cette question sera discutée. Enfin la loi sur la sécurité nationale de 2020 à Hong-Kong a porté un coup fatal aux cadres, un pays deux systèmes mis en place au moment de la rétrocession par le Royaume-Uni de Hong-Kong à la Chine en 1997. Le procès de 47 personnes accusées de subversion pour avoir organisé une élection primaire non officielle à Hong-Kong, en 2020, a commencé le mois dernier. Il vise à écraser la dissidence. La plupart de ces personnalités pro-démocratie sont détenus depuis 2 ans. Seuls 16 d'entre elles seront jugées alors que 31 personnes ont plaidé coupable et seront condamnés à l'issue du procès. Pékin s'est affranchi du respect de ses engagements internationaux, comme l'a dénoncé l'ONU et l'avait anticipé Josep Borrell ce procès le démontre. Est ce que l'Union européenne prévoit de prendre position. Sur ces procès politiques qui nous rappelle les procès staliniens et démontre que le concept qu'un pays 2 systèmes a disparu. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et enfin, la parole est à notre collègue Guillaume Chevrollier du groupe les républicains pour huit minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des Affaires européennes. Mes chers collègues. Le Conseil européen qui se tiendra les 23 et 24 mars prochain intervient dans un climat extrêmement compliqué pour l'Union européenne écartelée entre plusieurs crises distinctes, la première d'entre elles, et bien sûr la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dont nous fêtons le triste anniversaire. Une année pendant laquelle l'Europe n'a cessé de Tanguy face aux répercussions de ce conflit. Des répercussions humaines d'abord avec un bilan humain dramatique. Et des déplacements massifs de population. Je veux à ce titre saluer l'ensemble de nos collectivités locales nos élus, mais aussi nos concitoyens français comme je l'ai vu dans mon département de la Mayenne qui par pure solidarité ont permis à des familles de pouvoir être accueillis dans des conditions décentes sur notre territoire. Ce conflit a des conséquences militaires également pour la France et pour l'Europe avec l'envoi de matériel comme des canons Caesar. Pour la France et aussi des munitions. L'Union européenne devrait d'ailleurs fournir une aide de 2 milliards d'euros en munitions pour l'Ukraine, le double de ce qui était prévu. En mettant fin à la paix européenne si durement acquise. Cette guerre nous a conduit à nous interroger de façon lucide sur nos capacités militaires et les revoir au niveau national mais aussi au niveau européen. Quel est l'état actuel de notre coopération militaire avec nos voisins européens. Existe-t-il une ligne rouge à ne pas franchir dans l'aide apportée à l'Ukraine. Le prochain conseil européen va-t-il de nouveau débattre de sa boussole stratégique pour la, pour l'Europe de la défense. Ce conflit a engendré également une instabilité sur les marchés de l'énergie avec une augmentation vertigineuse des prix. Nous connaissons là aussi parfaitement bien les répercussions de ces prix de l'énergie sur nos collectivités locales sur toutes nos entreprises avec des factures insupportable pour beaucoup d'entre elles, je pense à nos artisans à nos commerçants. Couplé à un sous-investissement dans la filière nucléaire en France et l'arrêt de nombreux réacteurs. La France a échappé de peu à la catastrophe cet hiver mais qu'en sera-t-il l'année prochaine. Au niveau européen, notre politique d'investissements dans le nucléaire nous impose de réformer le marché européen de l'électricité. Découpler le prix de l'électricité. Les cours du gaz. Peut être. Le conflit avec la Russie et la suppression de l'approvisionnement en gaz russe a totalement changé la donne. Aujourd'hui, le mécanisme est devenu totalement inéquitable. Alors que le gaz ne contribue qu'à 7% de la production de notre électricité. La France doit peser de tout son poids dans les négociations à venir. À l'heure où nous relançons nos investissements dans le nucléaire. Peut-on espérer voir les négociations aboutir avant cet été. L'Union européenne est aussi tiraillée par la récente mise en place par les États-Unis de l'inflation réduction Act qui repose notamment sur un impressionnant paquet de subventions du gouvernement aérien américain à hauteur de 300 soit de 70 milliards de dollars pour stimuler le développement des énergies renouvelables. Ces mesures prises par les États-Unis constituent une véritable offensive économique. Et une volonté d'aller chercher en Europe des entreprises et leur technologie afin de les installer aux États-Unis en effet pour être éligibles à ces subventions. Les entreprises produire sur place. L'Union européenne doit réagir fermement risque de connaître une fuite des cerveaux et pire encore une fuite de notre savoir-faire technologique et industrielle. Les premières pistes d'une réponse européenne notamment via le Pacte Vert apparaissent mais semble néanmoins insuffisante. L'assouplissement des aides d'État permettra à la France d'investir davantage mais il aura comme conséquence de créer une distorsion au sein de l'Union européenne entre les pays membres, avec une forte capacité fiscale. Pour rappel, on estime que l'Europe aura besoin de 350 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an sur cette décennie pour atteindre son objectif de rémission de de réduction des émissions à l'horizon 2030 pour les seuls systèmes énergétiques. Néanmoins, la volonté de mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne ne peut être que saluée et encouragée pour 2 raisons écologiques et économiques. L'Union européenne a réalisé plus de 2100 milliards d'euros d'importation 2019 soit l'équivalent du PIB de la France. Des échanges intenses qui représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre européen. Cette mesure permettra de réduire cette empreinte carbone si importante à l'heure de la décarbonation de notre économie. Mais il constitue aussi une mesure de compétitivité économique avec cette taxe carbone Union européenne encourage la mise en place d'une concurrence loyale entre les entreprises européennes et les entreprises mondiales et une lutte contre la délocalisation de nos entreprises. Pouvez-vous Madame la Ministre de nous faire un état de la mise en place de cette taxe carbone et nous confirmer qu'elle sera bien effective en 2026. sans aucun doute l'empilement des réglementations ça. L'Union européenne qui pèsent sur nos entreprises et qui est devenu un des problèmes majeurs ces dernières années, 116 propositions de réglementation de la Commission européenne seraient en attente elle prévoit pour la seule année 2023, de présenter. 43 nouvelles initiatives. Madame la Ministre pensez en particulier à nos agriculteurs à ce secteur agricole si important pour notre souveraineté alimentaire si fortement fragilisée dans sa compétitivité. C'est une véritable surcharge réglementaire qui peut contribuer à faire peser sur nos entreprises des contraintes supplémentaires. Récemment encore dans cet hémicycle je rappeler combien les initiatives européennes en matière de RSE cette même et ceux si utile et nécessaire. Mais les les nouvelles initiatives c'est à craindre un choc de complexité en en élargissant l'obligation de diffusion d'informations sociales et environnementales. Un grand nombre d'entreprises européennes qui n'était jusqu'alors pas concernés notamment les PME. Peut-on espérer Madame la Ministre une Europe moins technocratique. Assistera-t-on cette année à la fin de la naïveté européenne à la fois militaire mais aussi économique, je le souhaite réellement il l'appelle de mes voeux. Je terminerai simplement cette intervention pour rappeler que nous sommes profondément européen. Eh bien évidemment tous attachés à l'Union européenne comme institution politique mais nous avons le devoir de nous réformer de nous adapter aux nouvelles réalités à un monde qui change, il y a une mondialisation qui notamment sur le plan environnemental a atteint ses limites se réformer. C'est la condition sine économe pour une Europe forte pour une Europe qui soit vraiment une Europe puissance face aux nombreuses menaces face au retour des des empires mais aussi face aux nombreux défis enthousiasmant du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent à madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Je pense que vous serez plus à l'aise. Sur le pupitre. Madame la ministre. Oui je pense que vous serez mieux là. Merci madame la présidente. Je recommence. Alors madame la présidente, monsieur le président, monsieur le rapporteur général. Mesdames, et messieurs les sénatrices et les sénateurs, vous m'avez. Je vous remercie d'abord pour vos interventions. et toutes les questions que vous m'avez posé je vais y tâcher d'y répondre le plus possible mais évidemment je vous prie de bien vouloir m'excuser. Le temps qui m'est imparti est restreint. Je sais que vous avez des. Une séance tôt demain matin. Je serais à votre disposition ainsi que mon cabinet. Si vous avez besoin de. Qui de réponses supplémentaires. J'ai commencé par l'Ukraine. Beaucoup d'entre vous. Monsieur le Président rate pas madame la sénatrice Guillotin. Le sénateur Gattolin madame la sénatrice mélo. Vous m'avez monsieur le rapporteur général Husson. Vous avez été nombreux à évoquer la guerre en Ukraine et effectivement les combats restent. Très intense. Alors la première question qui m'a été posée. Notre aide militaire à l'Ukraine et notamment les munitions et comme vous savez les 10. Question se poursuivent à Bruxelles. Sur les munitions les Ukrainiens en ont cruellement besoin la Russie tire environ 10.000 obus par jour. Une initiative de 2 milliards d'euros et proposé prélevés sur la Facilité européenne de paix pour accélérer la fourniture de munitions à l'Ukraine. Essentiellement du 155 millimètres pour être précise. Il y a un triple objectif. Le 1er d'encourager la cession des stocks en remboursant à hauteur de 1 milliard. Selon faites par les États membres à l'Ukraine. Faciliter les achats. Conjoints via l'Agence européenne de défense et puis renforcer les capacités de production de l'industrie européenne, notamment en utilisant le budget européen pour aider nos industriels à augmenter l'offre européenne Cette initiative devrait être validé lors du Conseil Affaires étrangères défense du 20 mars puis endossée au Conseil. Européen. Monsieur le sénateur, vous m'avez demandé s'il y avait une ligne rouge dans l'aide à fournir à l'Ukraine. Je crois que le président a été très clair sur le sujet. Rien n'est exclu mais nos choix doivent répondre à 3 exigences d'abord être efficace et utile immédiatement pour les Ukrainiens, ce qui n'est pas le cas comme vous savez de tous, de toutes les armes que nous leur passons. Ne pas contribuer à l'escalade et ne pas obérer nos propres capacités de défense

à mentionner les transferts forcés massif d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie et vous avez raison, ces transferts forcés sont absolument ignoble et et le Conseil européen s'est déjà emparée du sujet. Le dixième paquet de sanctions contre la Russie, adoptée le 25 février. A déjà permis de sanctionner quatre personnes responsables de la déportation et de l'adoption forcée d'enfants ukrainiens. Il s'agit de de responsables politiques dans des régions russes, le vice-1er ministre de la République du Bachkirie et le chef adjoint de l'oblast de Moscou. De la commissaire russe pour le droit pour les droits de l'homme ainsi que d'une responsable de fondation russes qui ont tous contribué à l'adoption illégale d'enfants ukrainiens par des citoyens russes. Évidemment nous n'hésiterons pas à renforcer ses sanctions. Monsieur le président. Hein monsieur sénateur qui autant vous m'avez également interrogé sur la Moldavie et madame la sénatrice Guillotin, excusez-moi. Il est tard je suis désolé. effectivement j'ai été la semaine dernière. Et je. Vous avez soulevé la question d'y aller, je ne peux efficace. Estimant que vous encourager. À aller apporter votre soutien à la Moldavie et à sa présidente. Maya Sandu. Il y a 3 thématiques principales que nous avons abordé la semaine dernière, notre coopération pour renforcer la démocratie, l'État de droit et la justice en Moldavie et vous savez comme la présidente s'est attaqué à la corruption dans son pays et la rénovation de la justice. Notre soutien à la société civile moldave. Notamment dans la continuité de l'aide d'urgence qui est apportée depuis l'an dernier et puis les préparatifs du 2ème, sommet de la CPE, le 1er juin Alzina qui sont effectivement très important pour. Pour la Moldavie. Donc je crois qu'il a des diplomatie parlementaire a vraiment un rôle très important à jouer et d'ailleurs c'est fréquemment le cas que dans les pays notamment des Balkans, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure la demande de soutien parlementaire est très très forte. Monsieur vice-président qui a dit que. Vous avez parlé de la Géorgie et j'ai eu l'occasion ce matin de recevoir la présidente de la commission des affaires européennes du Parlement géorgien. Vous avez rencontré également si mes informations sont bonnes. Le pays a 12 recommandations à mettre en oeuvre. Elle m'a fait part des progrès sur 11 d'entre eux le sujet polarisation de la vie politique de Morand un sujet difficile. De notre côté, nous avons salué le retrait du projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère puisqu'il n'était pas compatible avec le processus de rapprochement de la Géorgie avec l'Union européenne. Je crois qu'ils ont besoin de tous les soutiens et notamment techniques possibles en pour arriver à mettre en oeuvre les recommandations de façon qui soit satisfaisante et plus largement. Vous m'avez parlé de l'élargissement et des Balkans occidentaux et c'est un vrai sujet. De, d'arriver à fournir une assistance technique plus importantes. De façon à ne pas les laisser dans une chambre d'attente qui soit trop longue. Voilà pour l'Ukraine et le voisinage en ce qui concerne l'énergie, pardon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et notamment de. Répondre aux bonnes personnes donc monsieur le rapporteur général Husson mesdames et messieurs les sénatrices Berthet joli Chevrollier faire Nick. Vous m'avez interrogé. Mais oui, également. Guillotin mélo et Arnaud, pardon. Je crois que j'ai tout le monde hein. Vous m'avez. Interrogé en fait sur la compétitivité de l'Union européenne à travers l'énergie les questions sur l'énergie et sur les 9 Léchenne réduction Act. Ce que je crois, comme vous le. première, la première des raisons pour laquelle nous avons un fossé de compétitivité avec les États-Unis et d'autres régions. C'est bien le prix de l'énergie. Et dans ce cadre effectivement la réforme du marché de l'électricité est extrêmement importante et la France s'est mobilisée avec notamment le ministre Bruno Le Maire, la ministre Agnès Pannier-Runacher et tout le gouvernement depuis le début, pour protéger les consommateurs, lutter contre la volatilité des prix et puis donner de la visibilité à nos entreprises pour qu'elles puissent prendre leurs décisions d'investissement en Europe. Je crois qu'il faut reconnaître que la proposition de la Commission européenne est une base solide et large puisqu'elle inclut le nucléaire existant. elle va à la fois après vous réserver les avantages de l'intégration des échanges d'énergie en Europe mais elle nous apporte aussi. Des bénéfices concrets en matière de stabilité. Je disais il y avait va nous permettre de bénéficier de la compétitivité du parc. Nucléaire. Il y a à la fois les contrats à long terme que certains d'entre vous ont demandé à la fois ce qu'on appelle les contrats pour différence et les PPA qui permet de sécuriser les consommateurs comme les entreprises en incluant le nucléaire existant, de faire baisser les coûts, plus près des prix pardon plus près des coûts de production de notre parc nucléaire existant également. Et puis de fournir une certaine stabilité une prévisibilité qui est très importante pour nos entreprises. Notre objectif, c'est que cette réforme soit adoptée avant la fin de l'année nous aurons. Probablement des orientations en juin. Évidemment et je crois que le Parlement européen aussi en fait un sujet d'importance d'arriver à conclure de façon à pouvoir aller aux élections européennes. Avec cette réforme. Comme dans son bilan. Après les prix de l'énergie. Effectivement il y a la réponse. Avec le plan zéro émission nette.

Il y a plusieurs choses, d'abord un volet de propositions sur les marchés publics pour que tous les bons critères soient pris en compte dans l'attribution des contrats que ce soit la performance environnementale mais aussi la sécurité. Sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne. L'objectif étant que nos services publics ne soient pas assurés par des entreprises de pays tiers pour éviter toute dépendance. La 2ème chose c'est la mise en place d'une plateforme d'investissement pour mieux coordonner les financements disponibles et pour mobiliser toutes les ressources sur les secteurs stratégiques de façon rapide. J'entends monsieur le rapporteur général. Ce que vous dites sur la bureaucratie européenne, mais je peux vous assurer que le 3ème pilier de ce plan et la réduction des délais d'octroi de permis pour faciliter la réindustrialisation de de la France qui sera complété par le futur projet de loi industrie verte en France qui est porté par Bruno Lemaire. Nous voulons réduire la bureaucratie européenne et faire de la rapidité de nos procédures, un réel Avantage compétitif. Je ne dirais pas qu'il y a encore des progrès à faire, notamment dans cette. Proposition. La liste des technologies couverte doit être étendu pour intégrer le nucléaire puisque comme vous l'avez vu ce n'y est pas encore de même que la chaleur renouvelable. Et la biomasse. Il faut que le règlement prenne en compte tous les projets de décarbonation du secteur industriel. Alors comme je ne veux pas être trop long, je vais passer au Royaume-Uni. Comme le l'demandé madame la sénatrice Mélo. Messieurs les sénateurs gâteau Entre autres. Donc il y a effectivement eu l'accord dit de Windsor, le 27 février dernier, qui est une bonne chose puisque ils nous permettent d'avancer sur la mise en oeuvre du protocole nord-irlandais, il était assez simple, puisque vous m'avez demandé des détails pratiques, il y aura des produits destinés à rester sur le marché britannique et des produits qui iront sur le marché unique sur le marché britannique. Il y aura des tests aléatoires. Et pour ceux qui iront sur le marché unique des tests systématiques nous aurons un système de contrôle des données d'échanges commerciaux, de façon à détecter toute éventuelle fraude. Plus largement avec le Royaume-Uni, la ligne française n'a pas varié exigence maximale sur le respect des accords conclus dans le cadre du Brexit. Et ouverture maximale à travailler avec le Royaume-Uni, car nous n'étions pas à notre géographie. messieurs faire niquer Gattolin Arnaud et Chevrollier en ce qui concerne l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. La France est très clair et et le réaffirme, il faut garder cet objectif de 2035. D'abord parce que c'est un signal clair de notre mobilisation pour lutter contre l'urgence climatique. C'est donc nécessaire sur le plan écologique, mais c'est aussi nécessaire sur le plan industriel, nous l'avons dit. Aux producteurs de voitures, changer de direction ne, ne, n'est. Seraient tous nuisibles à la prévisibilité que nous voulons donner à toutes nos entreprises Donc c'est à la fois une décision écologique et industriel et puis elle nous permettra de renforcer notre indépendance énergétique. Je note aussi que la ministre de l'environnement allemande ne dit pas autre chose. Ce qui me donne beaucoup d'espoir pour sortir de cette situation malheureuse. Mais pas que de l'espoir. Monsieur, je vous assure du travail aussi. Monsieur les sénateurs Gattolin. Vous m'avez parlé de la visite du Premier ministre. Hongrois Viktor Orbán à Paris. L'objectif était clair, il était de rappeler. Que la Hongrie doit ratifier le Parlement hongrois. L'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Il est aussi de rappeler l'unité nécessaire, des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe des coopérations concrètes dans le cadre de la FCPE et le nécessaire renforcement de l'Europe de la défense. Enfin sur les travailleurs des plateformes. Il est vrai de dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Sous la présidence suédoise, vous saviez que le dernier conseil psycho n'avait pas été conclusive donc cette semaine il n'y a pas eu d'avancer les discussions vont se poursuivre. Et vous pouvez compter sur la France pour défendre une position constructive et équilibrée. Ce qui me donne l'occasion. De répéter que la commission n'exigent en rien une réforme des retraites. C'est une recommandation. Ce n'est pas un jalon du plan de relance. Ce qui est différent. Je suis sûr que vous en conviendrez. Et sur le DMA DSA comme vous savez, la mise en oeuvre est en train de se faire et les travaux du gouvernement se poursuive pour adapter les textes dans la législation et un projet de loi devrait vous être soumis à la fin du 1er semestre. Je vous remercie de votre attention de votre patience et de votre intérêt. Merci madame la ministre, hein. Pour conclure le débat. La parole est à monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Oui madame la présidente, madame, merci madame mamie. Merci cher collègue d'être. D'être resté si tard. Je sais que les uns et les autres. Depuis trois semaines, nos organismes nos nuits sont courtes. c'était vraiment obligatoire de, de faire ce. Ce débat près conseille à à cette date. En tout cas la conférence des présidents en avait décidé ainsi Madame la Ministre merci encore des réponses. Assez précise que vous avez pu porter mais vous, vous avez vu les questions étaient finalement assez groupé. Sur des sujets. Je l'ai dit déjà la dernière fois, je le redis, c'est la preuve que c'est vraiment redondant mais c'est finalement la la structuration et toutes les décisions qui sont prises autour de l'Ukraine bien sûr et de qui, de ce qui, de ce qui pourrait se passer. Je je je le dis très vite et sans rentrer dans le détail du propos de Thierry Breton, à nos côtés lundi soir. C'est vrai que la situation est vraiment dramatique. Elle est vraiment dramatique. Sur le plan humain, bien sûr, mais aussi sur le plan politique et géopolitique, donc. L'effort doit continuer à être à être reportée y mettre tous les moyens en tout cas je pense que. Ici, dans cette chambre vous auriez vous Le terme unanime et peut être très large mais en tout cas un un soutien très majeur. Madame la ministre, il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas évoqué est normal puisqu'ils n'interviendront pas dans le cas de ce conseil, mais il y a plusieurs sujets sur lesquels je voudrais ouvrir peut-être la suite de nos discussions. Dans, dans les semaines à venir. Parce que finalement on voit qu'il y a beaucoup d'opérations, ligne flèche une réduction Act, donc avec beaucoup d'engagement financier, probablement il y a bien sûr la guerre en Ukraine et donc un aspect budgétaire et financier non négligeable. Donc on doit avoir vraiment une réflexion est en tout cas. Avancer dans le travail De la révision du CFP du quad financier pluriannuel puisqu'on sait que sa révision. Viendra incessamment sous peu avec probablement à budget égal des, des lignes qui vont bouger. Au détriment de qui. Au détriment de quoi au profit de qui. Au profit de quoi. Je pense qu'il y a il y a vraiment la une une réflexion importante et puis le pacte de stabilité.

Vous ne me répondrez pas ce soir mais en tout cas j'ouvre sur les les prochaines sur les prochaines semaines. Merci en tout cas à tous je ne prolonge pas bonne soirée bonne nuit et à demain matin 9h. Merci. Mes chers collègues, nous en avons donc terminé avec ce débat si important et est fort intéressant. Je vais lever la séance prochaine séance demain jeudi 16 mars à 9h pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, la séance est levée. Bonne nuit cher collègue. Merci.